La séance est ouverte, le compte rendu analytique de la présente enseigne. Est distribué, il n'y a pas d'observation. Le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. Lors du jour appelle donc la discussion de la proposition de loi visant à à renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité aux fonctionnaires, présenté par monsieur Jean-Claude de recopier et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à madame Maryse Carrère du groupe RDSE, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, comme le reste de la société, l'administration est désormais confronté aux aspirations individuelles croissante et légitime de renouvellement professionnelle tout au long de la vie dans la durée, continue de s'allonger, entre 1946 et 2015, l'ex-l'espérance de vie a augmenté de 20 ans pour chaque sexe, passant de 59 à 79 ans pour les hommes et de 65 à 85 pour les femmes, l'allongement consécutif de la durée de leur carrière, un impact indéniable sur les projections professionnels des individus qu'ils évoluent dans le secteur privé ou dans le secteur public, les statistiques publiées sur le portail de la fonction publique, confirme cette intuition, on peut y lire que 40 pourcent des agents un situation de mobilité sont âgés de plus de 50 ans des dispositions législatives actuelles offrent en principe à tous les agents publics de grandes possibilités de mobilise. C'est entre administrations, mais aussi vers les organisations internationales, le secteur privé et un certaine nombre d'entités telles que les autorités administratives indépendantes. Elle leur permet également, dans des conditions particulières de se mettre en disponibilité afin d'exercer un mandat politique ou de donner la priorité à leur vie familiale, dans des conditions précises dans les faits, cependant, on constate que l'accès à la mobilité varie sensiblement selon la catégorie des agents, selon les données disponibles sur le site internet de la fonction publique, les agents de catégorie A Plus sont les plus mobiles

4 hôpitaux catégorie B et 5,7 pourcent des catégories C, cela peut s'expliquer de plusieurs manières : en 1er lieu la grande qualité des profils des agents de catégorie A, plus les rames particulièrement apte à valoriser leurs compétences dans l'ensemble des employes que notre société à offrir à l'absence de définition légale une problématique sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. On peut un effet considérer que les agents de catégorie A Plus sont ceux issus des écoles d'application les plus prestigieuses de la République, l'ENA, Polytechnique, les mines, les ponts et d'autres encore par leur prestige ces écoles attire d'excellents élèves qui pratiquent aussi parfois le cumul, c'est particulièrement vrai pour l'ENA où l'on trouve de nombreux anciens élèves des écoles normales supérieures ou de la Haute école de commerce. En France, où la théorie du signal se vérifie quotidien quotidiennement sur le marché de l'emploi, le profil du haut fonctionnaire ayant passé tous les filtres de la sélection républicaine est particulièrement recherchés. Cette importante mobilité peut également s'expliquer par des règles coutumières propres à certaines corps ou les départs seraient encouragés en raison des perspectives limitées de carrière pour des individus parvenu dès leur sortie d'école, à des niveaux hiérarchiques très élevé, les propositions du 1er comité interministériel de la transformation publiques tendent d'ailleurs à confirmer cette hypothèse puisqu'il est prévu que les élèves de l'ENA, sorti les mieux classés seront affectés au bout de 2 ans sur des postes consacrés à la mise en oeuvre des chantiers prioritaires du gouvernement d'administration centrale et dans l'administration territoriale, on peut lire cette proposition comme la volonté de satisfaire le besoin d'aventure des jeunes aux fonctionnaires et de mieux employer leur dynamisme sans remettre en cause leur place dans la guerre archi-décor puisqu'ils resteront à vie lié à leur administration d'affectation d'origine mais cela, cela remet également en question le besoin de recrutement des institutions concernées, comme vous nous en avaient informé Madame la rapporteur plusieurs de vos interlocuteurs ont insisté sur la crise d'attractivité que la haute fonction publique traverserez on observe pourtant que la sélectivité du concours externe de l'ENA reste supérieure à celle des écoles de commerce, plébiscité par le secteur privé, la rémunération actuelle apparaît comme un des facteurs principaux facteurs de découragement des agents de catégorie A Plus à construire toute leur carrière au service de l'administration, toutefois, parallèlement aux évolutions des aspirations individuelles des fonctionnaires que je viens de décrire. Les exigences éthiques de la société envers l'État se sont renforcées dès 1789 l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, prévoyez que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration au fil des siècles, ce principe est devenue plus effectif avec le renforcement de la publicité progressive des actes pris par l'administration, puis les premières lois de lutte contre les conflits d'intérêt et l'interdiction des rétrocommissions ou encore l'encadrement des paiements en espèces en parallèle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment la théorie des apparences a contribué à modifier le fonctionnement des juridictions administratives afin de lever toute suspicion de conflit d'intérêts possible entre la fonction juridictionnelle et la fonction de l'expertise juridique du Conseil d'État auprès du gouvernement ou encore enfin, afin de clarifier les rapports entre le rapporteur public et le reste de la formation de jugement, ce mouvement a irradié tous les pans de la société jusqu'aux lois instaurant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et renforçant les obligations déontologiques des fonctionnaires sous le gouvernement précédent. Ou, plus récemment encore, la loi pour la confiance dans l'action publique au cours de ces débats, plusieurs d'entre nous ont proposé de renforcer les dispositifs s'imposant aux fonctionnaires dont l'influence dans la conduite de la politique de la nation est déterminante, nos concitoyens doivent avoir à l'esprit qu'elle se manifeste à tous les stades de l'action publique au moment de l'Ebola Bora. De la loi, les administrations, sous l'autorité de leur directeur sont chargés de la préparation des projets de loi du gouvernement ensuite soumis pour avis aux membres du Conseil d'État pour avis sur la pertinence juridique des textes qui seront ensuite soumis au Parlement, une fois les lois adoptées les administrateurs civils sont ensuite chargés de rédiger les décrets d'application, sans lesquels les lois restent des lettres mortes, au-delà de l'élaboration des normes et aux fonctionnaires disposent également de rôle décisionnel important selon qu'qui soit chargé de conduire des négociations internationales au nom de la France, de régler des différends entre l'administration et les administrés d'engager des dépenses publiques, ou encore de prendre des décisions économiques substantielles leur décision ont le pouvoir de favoriser les intérêts des hommes ou des autres dans des circonstances plus confidentielles que celle de l'approcher procédure législative, les parlementaires faisant désormais l'objet de nombreux contrôles mais surtout dans des proportions plus importantes que les décisions prises par les agents de autre catégorie placés sous leur autorité, selon notre point de vue ses prérogatives considérables, justifie de soumettre aux fonctionnaires à des règles déontologiques propres plus exigeante que celle prévue pour l'ensemble des fonctionnaires depuis 2016, fort de ces constats, nous avons décidé de vous soumettre à cette proposition de loi dans l'esprit d'examiner toutes les pistes envisageables pour renforcer la prévention des conflits d'intérêts s'appliqua particulièrement aux fonctionnaires, il s'agit en 1er lieu de renforcer le contrôle effectué par la commission de déontologie en a modifié à la présidence afin de la prémunir contre les accusations de complaisance vis-à-vis de telle ou telle corps mais également de rendre effective l'automaticité des contrôles des allers-retours effectués par certaines aux fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé, d'instaurer un contrôle au moment de la réintégration après de mobilité et de renforcer le contrôle des agents destinés à prendre part au pouvoir des sanctions du. Zahir des API, nous sommes donc favorables à la publication des avis et à la fusion à terme de la commission de déontologie et de l'HATVP introduites très justement par la rapporteure et validé par la commission des lois. Le lien entre la perception d'un risque de conflit d'intérêt et la grande mobilité Déo fonctionnaires est très vite devenu évident aussi avant nous, eu la volonté de proposer un meilleur encadrement dans le temps de la mobilité, alors que l'étude que sont les énarques devenus. Suggérer que certains hauts fonctionnaires passent plus de la moitié de leur carrière dans le secteur privé, le 3ème axe découle directement du précédent si la mobilité mieux encadrer alors une éthique de responsabilité doit être développée au sein de l'administration afin de pousser les agents des désirable poursuivre le reste de leur carrière dans le secteur privé a démissionné, effectivement, il y a à honorer leur engagement vis-à-vis de la société en remboursant le coût de leur scolarité, le cas échéant, afin de restaurer l'attractivité de la carrière publique d'autres évolutions pourraient être envisagées sur le plan réglementaire qui avait été évoqué lors du débat organisé à l'initiative du groupe RDSE l'année dernière, réserver l'accès aux grands corps par la promotion interne et améliorer la formation professionnelle continue au sein de la fonction publique, auquel on peut à présent ajouté la revalorisation des traitements, ces derniers choix sont entre vos mains. Monsieur le ministre merci.

Monsieur le président, Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mais chers collègues en 1945 l'ordonnance relative à la formation au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires portant création de l'École nationale d'administration souligner le sentiment B. au de voir que la fonction publique entraîne un sentiment encore largement par partagé chez les agents publics qui concourent quotidiennement au fonctionnement de nos services publics et de nos institutions, lors des auditions que j'ai conduite à plusieurs témoignages ont illustré le dévouement de grand serviteur de la nation pour des traitements inférieures aux rémunérations des hauts cadres des entreprises aujourd'hui encore, ceux qui font le choix de rejoindre le secteur privé demeure minoritaire, y compris au sein des catégories supérieures de la fonction publique, où la part des départs vers le privé est tout de même beaucoup plus élevé, il en ressort que la question de la rémunération du haut fonctionnaire, demeure le noeud du problème, problème que l'on peut d'ailleurs étendre à d'autres catégories de la fonction publique, beaucoup de mes interlocuteurs ont présenté la mobilité comme un lieu, un levier d'attractivité vers la haute fonction publique, il nous a été dit que le recrutement traversait une crise pour autant à défaut de données en ce sens, on ne peut déplorer que le sentiment de baisse d'attractivité des carrières publiques à charge, à charge pour vous, Monsieur le Ministre d'objectiver ce sentiment, en outre, c'est un 2ème aspect des conclusions que je tire de mes auditions la perception du pantouflage est très variable selon la fonction exercée les administrations les plus favorables au passage vers le secteur privé sont souvent celles dont les activités sont le plus en lien avec l'écosystème, il s'agit pour eux d'accroître leur efficacité administrative en s'imprégnant des problématiques que rencontrent les acteurs économiques, la difficulté, dans ces cas-là, et de s'assurer que l'argent une fois retourner dans la dans l'administration, retrouve son partielle son impartialité vis-à-vis de l'entreprise qui l'a recruté constitue conclusion que je tire de mes auditions et la grande opacité qui entoure la notion de haute fonction publique et en 1er lieu son périmètre réel dès lors qu'il n'est nullement défini, il existe bien le terme de catégorie A mais selon les personnes interrogées, le nombre de personnes concernées varierait du simple au double, entre 12000 et 34000 personnes, excepté les maîtres de conférence, il en va de même concernant les données relatives à leur mobilité chaque corps, chaque administration recueille ou non des données sur la mobilité de ses membres, l'étude que sans les énarques devenus ne permet pas de retracer les mobilités vers le secteur privé des polytechniciens dépend des mines et d'autres encore, si elle a plus longtemps les protéger, je crains qu'aujourd'hui cette opacité ne décervelés haut fonctionnaire, à une époque où la transparence est requise, partout, il me semble indispensable, Monsieur le Ministre, que la DGA AFP se dote des moyens et des outils nécessaires pour disposer de données chiffrées sur la mobilité de c'est aux fonctionnaires si la mobilité des fonctionnaires aidés aux fonctionnaires, y compris vers le secteur privé me paraît indispensable, elle doit impérativement s'articuler avec le respect des principes déontologiques destiné à prévenir ou à sanctionner tout conflit d'intérêts dans le cadre de leur mission de service public, certaines situations peuvent produire des faits constatés constitutifs d'infractions pénales et se manifester tant dans l'exercice Parrón, agent de ses fonctions au sein du secteur public, qu'en cas de pantouflage, c'est-à-dire, c'est-à-dire lorsqu'un fonctionnaire souhaite quitter ses fonctions publiques pourrait occuper un poste dans le secteur privé, cet équilibre entre d'une part, favoriser la mobilité des fonctionnaires, et d'autre part, éviter les situations de Pampelune, l'intérêt est difficile à établir, c'est jusque-là le rôle de la commission de déontologie de la fonction publique, qui constitue le pivot de la prévention des conflits d'intérêts et des agents publics, alors que ses prérogatives ont été renforcés par la loi, déontologie des fonctionnaires du 20 avril 2016, force est de constater qu'elle fait toujours l'objet de nombreuses critiques, ce qui a motivé le dépôt de la proposition la plupart des personnes auditionnées ont reconnu que les dispositions actuelles présentent plusieurs défauts également constatée par nos collègues députés Fabiana Olivier Marlex les dispositifs relative recouvrement de la pantoufle ne sont guère opérationnelles, selon qu'ils interviennent après l'interruption de la scolarité où, après quelques années de service, le respect des règles de déontologie imposées depuis 2016 sont inégalement appliquée selon les ministères ou les administrations concernées, bien que la loi rendent la saisine de la commission de déontologie obligatoire, celle-ci ne dit pas, ne dispose pas des moyens de contrôler que tous les cas de mobilité entrant dans le Champ de l'article 25 oct et ont été soumis, l'activité de la commission de déontologie a également été critiquée en raison de la non-publication de ces avis et sa partialité a parfois été remises en cause. principe, le principe même de cohabitation de la commission de déontologie et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique n'est pas satisfaisant, je rappelle à ce titre que la HATVP est déjà chargé de collecter les déclarations de Patrimoine de certains hauts fonctionnaires dans ces conditions et souci soucieuse de remplir mon devoir de biche, activité qui évoquait Philippe Bas, j'ai été amené à proposer en tant que rapporteur pour la commission des lois désormais des amendements tant en attendant pas supprimer plusieurs articles du du groupe RDSE je les fais dans le souci de respecter au mieux la sensibilité des membres de la commission des lois, sur cette question. Il s'agit, il ne s'agit pas de schizophrénie, mais simplement de pensée complexe en conséquence si certains collègues regrettent la suppression de plusieurs articles de cette proposition de loi par la commission des lois, les dispositions restantes me paraissent importantes pour répondre à l'objectif que nous a signé cette proposition, une meilleure prévention des conflits d'intérêt dans la fonction publique et en particulier dans la haute fonction publique aujourd'hui, la commission de déontologie de la fonction publique est uniquement compétente lors donne des du départ de fonctionnaires d'un agent public vers le secteur privé dans ce cadre, elle apprécie la compatibilité des fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des 3 années précédentes avec celle qu'il exercerait au sein d'une entreprise du secteur concurrentiel. La commission des lois adoptées en en clarifiant la rédaction l'article 4 de la proposition de loi qui propose d'étendre la compétence de la commission, au retour d'un agent public dans la fonction publique après une partie de carrière et Fact dans un organisme privé à but lucratif, cette extension est apparu nécessaire, la prévention des conflits d'intérêt est indispensable aussi bien lors du départ d'un fonctionnaire dans le secteur privé recours, son retour dans le secteur public, dans ce cadre, la commission devrait à peu appréciée, la compatibilité de la nouvelle affectation du fonctionnaire dans la fonction publique avec les fonctions précédemment exercé dans le secteur concurrentiel, la commission des lois a également adopté l'article 5 en en clarifiant également la rédaction cet article propose d'étendre le contrôle de la commission de thé, anthologie de la fonction publique au recrutement des directeurs généraux et des secrétaires généraux des autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes, ce nouvel élargissement apparaît bienvenue, compte tenu des missions si des missions spécifiques exercées par ces autorités mission qui réclament de la part de leurs personnels comme des membres de leur collège, une neutralité totale dans l'exercice de leurs fonctions tout conflit d'intérêts ou soupçons de conflit d'intérêts pourrait nuire à la qualité des décisions rendues en outre, la commission des lois, introduit un article 4 bis qui visent à assurer la publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique, selon les mots qu'définirait elle-même concernant la suppression de l'article 6 qui proposait de plafonner à 5 ans la durée d'un détachement nos auditions ont souligné que le passage des fonctionnaires dans le secteur privé, son père désormais quasiment de façon quasi-exclusive par la voie d'une mise en disponibilité, faut-il prévoir un meilleur encadrement des mises à disponibilité, c'est une question dans le parlement devra se saisir enfin à l'article 7, la commission des lois adoptées l'institution d'une peine complémentaire obligatoire d'interdiction d'exercer une fonction publique pour les fonctionnaires coupables de crimes ou de certains délits, elle a en revanche supprimé du Champ de cette peine, les délits détachables de l'exercice d'une fonction publique qui font l'objet de sanctions pénales spécifique voilà monsieur le président, Monsieur le ministre mais, chers collègues, les modifications que la commission des lois adoptées, elles ne vise pas à bouleverser l'équilibre de la loi adoptée en 2016 n'étant au contraire à lui apporter des compléments utiles, je vous remercie de votre attention. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des Comptes publics. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission Madame le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons touche à une exigence la déontologie qui est consubstantielle à l'action publique, la déontologie, entendu comme la connaissance de ce qui est juste et convenable, rapporté à l'activité professionnelle participe en effet directement à la légitimité de l'action publique auprès de nos concitoyens, c'est exigence, imposent aux responsables politiques, mais elle doit également être au coeur de l'action des agents publics et plus particulièrement de ceux d'entre qui exercent les responsabilités les plus importantes et mettent en oeuvre les orientations arrêtées par le pouvoir politique, il ne peut y avoir de confiance publique que si les citoyens ont la conviction que ce qui la souveraineté délégués agissent au service de l'intérêt général c'est exigence de probité d'intégrité, d'impartialité n'est pas nouvelle pour notre pays, c'est en effet lui 9 qui, le 1er exigea des officiers placés sous son autorité qu'il réforme tout abus moral et politique, dans son ordonnance de 1954 tout au long de notre histoire, nous sommes collectivement, interrogé sur les obligations des fonctionnaires sur ce sentiment D de voir que la fonction publique entraîne pour eux 30, reprend les termes de l'ordonnance 9 octobre 1945 qui a conduit en particulier à la création de l'École nationale d'administration c'est exigence s'est toutefois considérablement renforcée ces dernières années alors que les attentes en matière de transparence et des gants d'exemplarité se sont accrues, la plus grande porosité, la plus grande mobilité professionnelle entre le secteur public et le secteur privé l'expliquent en partie. Ne nous y trompons pas, cette mobilité est une source d'enrichissement pour les agents publics pour le service public et pour la société dans son ensemble, les allers-retours professionnels entre le service public et le secteur privé favorise en effet pleinement la respiration et la créativité dans notre société a besoin, c'est tout le sens de la démarche engagée par le gouvernement dans le cas du programme Action publique 2022 afin de décloisonner le déroulement des carrières entre l'emploi public et l'emploi privé, par conséquent, s'il faut sanctionner efficacement les manquements aux règles ontologique, il faut éviter de créer des règles qui procéderait d'une suspicion généralisée à l'égard des agents publics et paralyserait de façon disproportionnée, efficacité de l'action publique c'est équilibré a précisément été consacrée à l'adoption de la loi du 20 avril 2016 relatives à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a emporté la plus importante réforme du statut général de la fonction publique en matière déontologique depuis 1983 comme vous le savez, cette loi rappelle les valeurs essentielles du service public qui sont portés par les agents publics elle défini organisme les mécanismes relatifs aux conflits d'intérêts et là sur une large diffusion d'une culture déontologique auprès des agents publics car la déontologie et moi faire d'interdire que de valeurs et de principes positif qui doivent être mises en Oeuvres de façon préventive, je ne reviendrai pas sur les dispositifs de prévention des conflits d'intérêts, mis en place par cette loi 2016 que vous connaissez parfaitement et dans le récent rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale relative relatif pardon à la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts, dresse l'inventaire je me permettrais simplement de rappeler plus emblématique d'entre eux, d'abord l'extension des compétences de la commission déontologie de la fonction publique qui contrôlent désormais systématiquement les départs, le secteur privé de tous les agents publics ensuite un encadrement plus strict des cumuls d'activité entre l'emploi public et une activité privée accessoires, la mise en place de référent déontologue dans les 3 versants de la fonction publique, afin que tout agent public dispose d'un interlocuteur clairement identifié sur ces questions, et enfin la mise en place d'un statut protecteur pour les lanceurs d'alerte, ces dispositions qui concernent l'ensemble des agents publics ont été complétées par des mécanismes de prévention des conflits d'intérêts spécifiques pour les emplois les plus sensibles des 3 versants de la fonction publique, certains employes sont ainsi soumis contenu, leur niveau hiérarchique ou la nature des fonctions exercées à des obligations déclaratives nouvelle les agents qui occupent ces emplois sont ainsi tenu du du de déclarer leurs intérêts, leur situation patrimoniale de confier à des tiers des mandats pour la gestion de leurs instruments financiers pour la seule fonction publique d'État, ce sont désormais près de 4500 emplois qui sont soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts et de 500 emplois pour la déclaration de de situation patrimoniale, s'agissant des postes les plus importants de l'administration, c'est-à-dire ceux à la décision du gouvernement comme par exemple les directeurs d'administration centrale, les secrétaires généraux de ministères la nomination sur ces emplois est également subordonnée à la transmission d'une déclaration d'intérêts et d'une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, l'articulation de tous ces dispositifs permet de prévenir de façon équilibrée la survenance de conflit d'intérêts à la sortie de l'emploi public vers le secteur privé, mais aussi lors du retour des agents concernés dans l'emploi public, qu'il me soit permis à nouveau de souligner que ce contrôle sur les emplois les plus exposés à la sortie, comme à l'entrée concerne tous les agents publics, fonctionnaires ou non, est-il aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin et de modifier comme vous le proposez, avec cette proposition de loi les dispositifs existants, ce n'est pas la position du gouvernement, non pas parce que le gouvernement ne partagent pas le même souci que le Sénat, quant aux exigences d'exemplarité et de probité attaché l'emploi public mais parce que les règles déontologiques existantes ont procédé de la volonté de construire un dispositif équilibré et qu'elle commence tout juste à être déployés certains des décrets d'application de la loi du 20 avril 2016, qui a été cité par madame la rapporteur et non des moindres, sont entrées en vigueur depuis moins d'une année, nous pouvons très difficilement juger aujourd'hui avec tout le recul nécessaire, de la nécessité de compléter notre corpus législatif en matière d'anthologie des agents publics, il nous faut avant tout désormais faire appliquer et faire vivre ses règles nouvelles : la réforme du législatif envisagée par le Sénat par cette proposition de loi nous semble donc aujourd'hui prématuré des adaptations seront sans doute ultérieurement nécessaires, notamment celles qui seront de nature à assurer tout en les encadrant la fluidité et le décloisonnement des carrières entre l'emploi public et l'emploi privé, à cet égard le gouvernement partage pleinement les conclusions du jeu les conclusions, pardon du récent rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, relatif à la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts, il s'agit moins de réviser le dispositif législatif que d'envisager son ajustement et le gouvernement, il restera particulièrement vigilants, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Madame la rapporteure promouvoir et veiller au respect de la déontologie au sein de l'administration est une condition essentielle à la pérennité du pacte républicain et la légitimité de l'action des pouvoirs publics, le gouvernement considère que le cadre législatif tels qu'ils existent et de nature à répondre à ces exigences d'éventuels ajustements pourraient intervenir, c'est sous réserve que les effets des obligations déontologiques, récemment mis en place était pleinement déployer évaluer, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons souscrire à la présente à la proposition de loi que vous nous avez merci. Dans la suite de Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour l'union centriste, il a 8 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois Madame le rapporteur madame l'auteur mais, chers collègues, le texte que nous examinons, aujourd'hui, est un texte que je qualifie volontiers de pragmatique, je tiens d'ailleurs à saluer, dans cette perspective, le travail de notre collègue Josiane Costes rapporteur qui a dû affronter de nombreuses résistance et réticence au changement, un texte pragmatique donc car nécessaire. Car si les fonctionnaires demeurent essentiels à l'organisation de notre pays, et si nous sommes pour le principe de mieux contrôler les pratiques en vigueur et pour la surveillance accrue des conflits d'intérêts éventuels nous demeurons tout de même vigilants à ce que la cela ne soit pas l'occasion de donner satisfaction à ceux qui cherchent à tout prix des boucs émissaires et nous, mes chers collègues, qui vivons parfois les affres de l'antiparlementarisme, nous devons être particulièrement vigilants sur ce point. Ce texte n'est plus que nécessaire de par son crâne caractère préambule est, en effet, les annonces du gouvernement, Monsieur le Ministre, sur le programme d'action publique 2022 on fait couler beaucoup d'encre, il est désormais nécessaire, est certain que nous aurons dans les mois à venir, à débattre d'une réforme globale du statut de fonctionnaire, donc nous aurons l'occasion de nous revoir et d'en reparler ici même. Avec l'annonce de ce programme le 1er ministre Édouard Philippe accompagné. De Gérald Darmanin, ministre de l'action et des Comptes publics et de vous-même Monsieur le le secrétaire d'État, vous avez dévoilé les 4 piliers sur lesquels la réforme de la fonction publique devrait reposer il reviendrait aujourd'hui que sur un des seuls. Point qui nous concerne directement et qui concerne l'objet de cette proposition de loi, le gouvernement prévoit, selon ses mots, de banaliser le recours aux contractuels dans la fonction publique, si l'objectif principal est de contourner le statut de fonctionnaire, j'ai comme trop rigide, le gouvernement invoque aussi pour justifier ce recours contractuels le besoin d'assurer la mobilité de l'ensemble des fonctionnaires et ne sont en effet chaque année que 4 pourcent à changer de poste, plus encore, il y a disparité flagrante entre les différents corps de l'État et surtout entre les différentes catégories de fonctionnaires, de fait, très haut fonctionnaires les fameuses catégories A jouissent de possibilités que n'ont pas les autres catégories, là où il les aller-retour avec le privé sont largement et facilement possible pour les uns, il n'y a que le contrôle strict et encadrement lourd pour pour les autres, au regard de la fonction publique dans son ensemble et hauts fonctionnaires ont une mob mobilité sans égal, c'est du reste ce qui justifie que cette proposition de loi s'intéresse particulièrement aussi aussi essentielle soit cette mobilité, il ne faut pas avoir peur de dire il y a des abus qui sont honteuses lorsqu'on sert l'État et constituent autant d'affront pour les corps auquel ces fonctionnaires appartiennent oui nous devons lutter contre les abus, car il dessert la fonction publique ternissent l'image du service public pousse non ses concitoyens à la défiance mais vous me méprenez pas sur mes propos, il ne s'agit pas ici de couvrir d'opprobre, ce qui, aussi, au service de l'État et de nos concitoyens remplissent chaque jour des fonctions éminemment importante censée aux fonctionnaires, notre service public ne serait pas, il s'agit donc de dénoncer ici les situations s'est singulièrement anormal que nous devrions ne plus tolérer j'ai évoqué tout à l'heure à la Mobilité, Mobilité sans égal pour les fonctionnaires par rapport aux autres catégories non troppo pas là non plus sur les conséquences de ce qu'on a on appelle familièrement le pantouflage, la mobilité est un élément essentiel du fonctionnement des grands corps de l'État en renouvelant des effectifs peu changeant, elle permet de placer les personnes les plus compétentes au postes les plus adéquats en cela la mobilité est saine et mérite d'être encouragée et cela sans tabou l'objet d'une OPA, ici, je le répète, de supprimer ou de porter atteinte à cette possibilité d'aller et de venir entre le public et le privé, mais j'en ai invité seulement les dérives plus encore cette mobilité permet de répondre aux besoins d'administration, de fait, il y a aujourd'hui un besoin croissant d'expertise technique l'efficacité d'une administration ou d'une autorité publique dépendant aussi et surtout du degré de connaissance des secteurs sur lesquels travaille, prenons l'exemple de l'autorité des maraîchers financier, l'État n'a que peu d'expertise particulière en la matière et ses fonctionnaires ne sont pas ou peu formés à ces problématiques l'essentiel du secteur étant privé, l'expérience de certains fonctionnaires, dans les entreprises privées depuis leur retour dans leur leur administration entraîne de fait un gars en expertise comment expérience un gain précieux puisque leur administration ne peut-être au niveau des secteurs qui influence voir elle réglemente qu'en connaissant les rouages propres à ces derniers, force est de constater que le pantouflage, si on peut le qualifier ainsi participent à cette connaissance, bien au-delà de ces exemples particuliers en plus de participer à l'expertise nécessaire dans les faire de l'administration, il convient aussi de rappeler que la mobilité d'une pratique encadrée : contrairement à ce que certains laissent entendre, tout n'est pas permis le code pénal prévoit en effet un délit de prise illégale d'intérêts dans son article 432 13 de plus, la commission de déontologie visés par la présente proposition de loi est d'ores et déjà chargé de vérifier qu'un agent de la fonction publique est légitime pour occuper des emplois privés auquel il postule malgré ces garde-fous, il y a, j'ai déjà dit des abus et pour nous, ils sont de 2 types. Le premier abus et celui qui concerne une minorité de fonctionnaires mais qui consiste dans l'Euro, non respect de l'engagement décennal qui incombe aux élèves de l'École nationale de Miss ration de l'École polytechnique et de l'École normale supérieure, le fonctionnaire qui élève vous voyez ces frais de scolarité, pris en charge par l'État se doit les rembourser s'il quittait l'immigration prématurément ses écoles dans les concours d'entrée, figurent parmi les plus difficiles de notre pays n'ont pas vocation à nos yeux à former des cadres d'entreprises privées, ces écoles sont créées pour démocratiser l'accès du plus grand nombre à la haute fonction publique, il ne faut pas que cet objectif initial se perdent mais bon type d'abus bien plus graves concernent des conflits d'intérêts auxquels peuvent être confrontés Les fonctionnaires vous n'êtes pas mes chers collègues, sans connaître la théorie de la capture qui décrit schématiquement comment les moyens de réglementation et le pouvoir Cities de l'État peuvent être utilisés orientés afin de desservir les intérêts privés avec la notion de pantouflage, nous nous rapprochons de cette théorie des genres Stiegler effectivement un fonctionnaire peut être tenté de favoriser l'entreprise en vue d'un poste futur ou ensuite, une fois de retour dans l'administration, au nom de relations professionnelles passées ces situations ne devrait pas se produire ne devrait plus se produire, c'est pourquoi nous ne sommes pas par principe opposée à la présente proposition de loi, ou du moins aux objectifs qu'elle poursuit ses propositions de loi n'aborde que l'espèce unique de la prévention des conflits d'intérêts, il est vrai que la commission de déontologie de la fonction publique doit avoir les moyens de jouer pleinement son rôle qui lui était destinée, lors de sa création en 1993 mais ce n'est pas là le seul moyen que nous avons pour contrôler le pantouflage et prévenir les conflits d'intérêts, il eût peut-être été plus constructif de réfléchir à un statut de la haute fonction publique avant que le gouvernement nous impose sa vision, plutôt que de ne se concentrer que sur les modalités de contrôle des amendements vont en ce sens, je pense que nous en reparlerons dans les minutes qui viennent, la confiance dans l'État et dans la fonction publique passe nécessairement par la prévention des conflits d'intérêts, mais trop souvent et à tort, les fonctionnaires sont désignés comme responsables des problèmes du pays, bien placé pour l'entendre pour en être parfois nous-mêmes parlementaires la vie les nous appelons donc de de nouvelles réforme globale de leur statut, incluant la reconnaissance statutaire d'une fonction publique de catégorie A plus tout en renforçant la déontologie de l'administration, c'est par là que passera la main des rations des services publics et le retour de la confiance des citoyens dans leurs administrations merci. La parole est maintenant à monsieur Jacques Bigot pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la commission des lois Madame la rapporteure, chers collègues, auteur avec votre groupe de ce projet de loi. Notre groupe est à l'égard de ce projet de loi extrêmement réservé, non pas sur la question de la lutte de la prévention contre les conflits d'intérêts, mais sur l'opportunité aujourd'hui de rajouter une loi à la loi. Je pense que nous devrions et on aura l'occasion souvent de dire nous inspirer fortement de ce que le Conseil d'État, monsieur le ministre vient de dire à votre gouvernement à propos de la loi des des mesures relatif à l'asile en disant une loi a été faite en mars 2016, vous n'avez pas eu le temps d'examiner comment elle fonctionne déjà vous voulez en faire une autre. J'ai bien noté effectivement que la proposition était de renforcer de rajouter des points mais a-t-on fait suffisamment le tour des difficultés de l'application de la loi de 1900 pour dire aujourd'hui il faut aller plus loin. Compléter, renforcer ce n'est pas Madame, rapporteur complètement votre sentiment et vous avez d'ailleurs fortement nuancer l'esprit de cette loi, je crois que sur ces sujets, il faut voir comment les textes sont appliquées, comment ils sont ressentis comment ils peuvent aller, c'est d'ailleurs aussi cette précipitation, monsieur le ministre, que vous avez en un autre temps de votre vie politique au mois de juillet dernier, lors ce que le nouveau gouvernement dont vous ne. J'ai pas encore membre s'est précipité pour faire une loi relatif au aux élus et vous-même vous aviez soutenu une motion de renvoi en commission, en disant : ce texte, c'est trop rapide, on n'a pas le temps de l'examiner vous Baader fait le griefs à la commission des lois de l'Assemblée, d'avoir exclu les propositions d'articles que nous avions fait sur la question des conflits d'intérêt dans la fonction publique, ça veut bien dire Michel reconnaît qu'il est indispensable sur ces sujets que nous prenons le temps de la réflexion ce que fait l'Assemblée nationale, avec un rapport d'information et, à partir de là, d'un certain nombre de débats pour voir si les choses ne fonctionnent pas, parce que le vrai sujet de la déontologie, c'est que la déontologie appartient corps social ce corps social, c'est celui de la fonction publique, nous avons fait le choix en 2013 de laisser ce corps social s'occuper de la paix ontologie les fonctionnaires. Y compris dans ces départs, avec notamment la Commission déontologie mise en place auprès du 1er ministre il nous faut voir si cette déontologie est appliquée la déontologie peut avoir le danger de n'être que l'exercice d'un corps social et elle ne se fait pas forcément dans la transparence et il peut avoir de la part de nos concitoyens devrait révéler une revendication de dire mais nous avons besoin de transparence et donc. La commission interne à une administration ne nous suffit pas, on veut qu'il y avait une haute autorité qui lié un organisme particulier qui soit indépendant qui puisse se prononcer, mais il ne faut à mon avis pas le faire dans la précipitation, il faut d'abord s'assurer que la haute fonction publique n'est pas capable elles-mêmes de gérer la question, le sujet reste éminemment compliqué éminemment compliqué parce que extrêmement délicat, j'entends que l'on dit très fortement, y compris l'actuel président de la République peut comprendre puisqu'il il a fait aussi des voyages hors d'or de la haute fonction. Public dont il est membre, a dit lui-même, c'est une richesse. Que de pouvoir à un moment donné, partir dans le privé et revenir dans le public. Certes, c'est une richesse, c'est d'ailleurs souvent aussi un enrichissement personnel, il ne faut pas le nier. ça peut être une chasse en terme de formation mais lorsque l'on voit, et je cite là le rapport de l'Assemblée nationale, lorsqu'on constate que l'essentiel des mouvements dans la haute fonction publique et dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, qui vont dans le secteur privé ou parmi les membres de l'Inspection générale des finances, peut se poser la question. On pourra se poser la question de dire est-ce que cela est possible. Nos grandes écoles sont là pour former, nous dit-on, l'élite de la nation, celle dont un certain nombre de nos concitoyens pensent peut-être, aujourd'hui, qu'elle gouverne plus la France. Que les élus eux-mêmes. Et encore moins les parlementaires auxquelles on a envie, par les réformes constitutionnelles en on vu encore du pouvoir. à partir de là, il faut un jour oser poser la question de dire mais est-ce que l'or, ce que l'on choisit de faire ces grandes écoles qui est destiné à la fonction publique. Est ce qu'on ne pourra pas rester d'abord dans la fonction publique mais si choisir à l'âge de 20 ans ou de 21 ans, de rentrer dans la fonction publique, c'est pour avoir un excellent diplôme qui vous permet d'être engagé ailleurs Eddy gagner très bien sa vie, c'est un vrai sujet, c'est au-delà de la notion de conflit d'intérêts. Et donc ce sujet, il faudra bien aussi pouvoir l'aborder parce que franchement je tiens tous, je cite toujours ce rapport, quand on voit que, en 2016, le directeur général du Trésor a rejoint comme manager de partenaires, un fonds d'investissement, on peut se poser la question de qu'est-ce que cela apporte-t-il à à la richesse de la fonction publique, est ce que ceci est tout à fait normal parce que si on l'a recruté, c'est bien évidemment en raison des compétences et de la connaissance qu'ils pouvaient avoir les portes ouvertes, les réseaux du mode de fonctionnement. Ce n'est pas ce que vous allez régler par cette proposition de loi. Vous allez à la marge, même si on reprend des amendements etc accompagné un peu ce qui s'est fait dans les textes précédents. Mais sur les conflits d'intérêts, on a déjà suffisamment de textes qui permet de sanctionner, on a suffisamment de choses et la déontologie, c'est d'abord un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui aujourd'hui peut-être dans la haute fonction publique n'apparaît pas suffisant. C'est peut-être cet état d'esprit qu'il faut redonner, en disant, comme vous l'avez dit, chers collègues, tout à l'heure, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que de pouvoir quitter un temps la fonction publique mais à mes yeux, c'est pour acquérir une expérience dans le privé qui va nourrir la haute fonction publique et pas nécessairement pour satisfaire les intérêts d'une carrière strictement personnel, ces mouvements-là sont utiles ces mouvements-là peuvent entraîner des conflits d'intérêts. Mais si dès leur formation. Léo fonctionnaires comme tous les fonctionnaires ont le sens de la fonction publique ont le sens de la déontologie, il n'y a pas bras, pas besoin de rajouter aux textes pénaux que nous avons déjà. C'est des états d'esprit qu'il faut nourrir, je ne suis pas sûr que le législateur, en rajoutant des articles ou des articles et en rendant les lois, comme l'a dit le Conseil d'État, à un moment donné, incompréhensible et il ne inapplicable, que l'on réussit. Dans l'objectif que l'on veut donner cette pour cette raison que notre groupe est très réservé par rapport à cette proposition, mais que sur le fond, nous attendons de voir ce qu'il pourra en rester parce que nous savons désormais, madame la rapporteur qu'il restera finalement.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président, la commission des lois Madame le rapporteur, mes chers collègues, notre pays peut compter sur une fonction publique de grande qualité qui s'inscrit dans une tradition ancienne de probité je souhaite leur particulièrement à cette tribune en souligner l'excellence. Cette proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts, aux fonctionnaires, dans le cas de leur mobilité dans le secteur privé ne relève donc pas d'une quelconque culture du soupçon d'autant plus que la déontologie et l'encadrement des conflits d'intérêts des fonctionnaires sont loin d'être des questions contemporaines. Les évolutions législatives récentes ne constitue qu'une étape assurément majeur d'un processus ancien l'émergence de principes déontologiques et d'un point de vue historique concomitante de l'apparition d'une catégorie d'agents spécialisés au service de la couronne à titre d'exemple, l'ordonnance de Saint-Louis en 1254 sur la réforme de l'administration et de la police du royaume consacrait déjà le principe d'intégrité des agents publics de nos jours la mobilité des fonctionnaires constituent un véritable outil de valorisation des carrières et des compétences, pour cette raison, elle doit être encouragé, d'autant plus que la France souffre d'un manque d'attractivité, parallèlement, il est important de demeurer vigilant quant au risque de conflit d'intérêts qui peuvent survenir en cas de pantouflage, l'équilibre entre la double nécessité de favoriser la mobilité des fonctionnaires et d'éviter les situations de conflit d'intérêts, doit être recherchée si les dispositifs légal actuel en matière de déontologie est abouti grâce aux dernières évolutions notamment il peut toutefois faire l'objet d'ajustements opérationnels, c'est ce qui explique les initiatives déjà prises par le Sénat et le dépôt par monsieur Jean-Claude Rech et plusieurs de nos collègues de cette proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité aux fonctionnaires. Si je souscris à l'objectif d'une prévention renforcée des conflits d'intérêts, ce texte appelle néanmoins un certain nombre de remarques tout d'abord, il apparaît difficile de quantifier la mobilité des fonctionnaires au secteur privé en raison à la fois de l'absence de données et de la définition de la haute fonction publique, ensuite on peut regretter que je texte arrive en examen alors que la loi du 20 avril 2016 n'est pleinement applicable que depuis le 1er février 2017, date d'entrée en vigueur des derniers décrets d'application, plusieurs dispositions de la proposition de loi soulève des questions Julie juridico-pratique qui risquerait de réduire l'attractivité de la fonction publique, sans pour autant permettre d'atteindre efficacement l'objectif recherché, telle le cas des articles 1er 2 3 et 6 que la commission des lois à supprimer à l'initiative du rapporteur. La commission a également modifié les articles 4 5 et 7 pour en affiner le périmètre d'application ou pour clarifier la rédaction, elle a enfin introduit un article 4 bis pendant à rendre obligatoire la publication des avis de la commission de déontologie de la fonction publique, selon les modalités que celle-ci fixerait je souhaite m'attarder sur cette disposition Kara question de la transparence est ici centrale cette initiative répond à la préoccupation des administrations qui regrette la méconnaissance des avis de la commission d'déontologie n'en étant pas destinataire par ailleurs cette publicité permettra de s'aligner sur les pratiques existant par exemple au Conseil d'État où les avis du collège de déontologie font l'objet d'une publication il n'Extenso aidés leurs délibérations sur le site internet où ils sentent anonymisés, enfin, je regrette que la transformation de la commission de déontologie en autorité indépendante n'ait pas été retenu plusieurs rapports relatifs à la déontologie dans la fonction publique dans le récent rapport des députés Matra ses Marlex préconise une clarification du positionnement institutionnel de la commission de déontologie qui est pour l'heure, placé auprès du 1er ministre l'exigence d'indépendance inhérente à ces travaux et le fait que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique soit devenu une autorité administrative indépendante en 2013 plaide pour ce changement de statut, j'ai donc déposé un amendement avec mes collègues du groupe des Indépendants visant à ériger la commission de déontologie de la fonction publique en autorité administrative indépendante, serait un 1er pas vers une fusion avec la Haute autorité de la transparence répondant Timsit à un souci de clarification et de simplification du cadre déontologique dans la sphère publique. Avant de conclure : je souhaite saluer l'objectivité et l'impartialité du rapporteur Josiane Costes qui a guidé l'ensemble des travaux, monsieur le Ministre, mes chers collègues, si de nombreuses suppressions d'articles ont été opérées au cours de l'examen par la commission des lois, en revanche, certaines avancées ne sont pas négligeables, comme la publication des avis de la commission d'déontologie ou encore l'extension de son contrôle au recrutement des secrétaires généraux et directeurs généraux des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes ainsi que vis-à-vis des fonctionnaires, réintégrant le secteur public, après un passage dans le secteur privé raison, pour ces raisons, le groupe des Indépendants votera en faveur de ce texte, je vous remercie.

Oui merci monsieur le président, Monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des lois, le rapporteur je salue aussi l'ensemble des collègues et naturellement les auteurs de cette proposition de loi concernant la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des qu'aux fonctionnaires, il s'agit là d'un sujet important et les quelques minutes que dont je dispose, je pense que là, c'est un sujet qui mérite aussi une attention toute particulière, c'est pour ça par rapport, je me permets de faire un peu le le rapprochement de cette proposition de loi par rapport test qu'on avait abordé l'été dernier, c'était dur, jusqu'au 4 août devant Madame le le le garde des Sceaux, sur la transparence de la vie politique, alors c'était pour les élus, élus, parlementaires, la réserve parlementaire, on avait évoqué beaucoup l'éthique, la morale, la transparence, donc on peut aussi faire le parallèle, donc je remercie vraiment l'auteur les auteurs au niveau du groupe rde qui se sont penchés aussi sur ce sujet important

ça date de la complexité, je dirais, parce que dans le fond, l'attractivité de nos fonctions publiques et on peut raisonner naturellement sur l'aux 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, avec l'ensemble des ministères, fonction publique hospitalière Fonction publique territoriale, la mobilité,

beaucoup d'exemples, l'a été évoquée naturellement par l'auteur de la proposition de loi, le problème d'attractivité de la fonction publique d'État, c'est non Fonction publique et c'est aussi des sujets qui ne sont pas simple du tout, alors, les autorités indépendantes ont été cités, la Haute autorité de la transparence de la vie publique, les fonctionnaires comme nous les parlementaires, un certain nombre aussi de l'UE, donc ça touche aussi beaucoup de de personnes pour la déclaration de Patrimoine, déclaration de conflits d'intérêts, je crois que, à ce niveau-là, les règles de déontologie aux fonctionnaires sont aussi essentiels ça été rappelé les valeurs, l'éthique, la morale avec une instance que vous avez cité la commission de déontologie de la fonction publique pour redéfinir aussi les les moyens les règles qui peut varier aussi d'un secteur à l'autre et vous avez ras appelé naturellement le dévouement de l'ensemble des serviteurs de de l'État, mais je l'associe aussi à nos 3 fonctions publiques, se pose aussi le problème de rémunération du liés aux fonctionnaires et naturellement le sentiment de baisse d'actes d'attractivité, c'est vrai, on peut faire le lien entre le public et le privé, et c'est un sujet aussi qui n'est pas simplement parce que je témoigne modestement, avec mes collègues de la commission des finances, quand on examine, on a examiné la la loi de finances pour 2018, regardez les moyens humains et d'une mission à l'autre ministère après ministère, on voit aussi l'importance des différentes catégories de serviteurs de l'État et de l'ensemble de nos fonctions publiques mais également la catégorie A

à tous les niveaux on peut ajouter naturellement l'ensemble des des ministères, y compris la défense, la sécurité intérieure, je crois à tous, à tous les niveaux et les chiffres ont été donnés 12000 à 34000 personnels madame le rapporteur, les inciter même on pourrait atteindre son 1000 si on ajoute les maîtres de conférence, donc je crois que c'est aussi des cirques, on doit prendre en compte et naturellement la mission de service public, l'intérêt général, la déontologie, c'est l'été rappelé : Monsieur le Ministre, vous avez insisté particulièrement sur les notions de confiance de probité d'intégrité qui sont les valeurs essentielles, je crois que ça vaut à tous les niveaux, c'est pour ça que je me suis permis aux nouvelles un petit peu le lien que nous avions fait par rapport à la transparence de la vie politique et on peut le faire d'un côté, les élus, les parlementaires l'ensemble des élus, puis de l'autre côté, Valéo aux fonctionnaires c'est et c'était donc sa tête ça réellement au moins le mérite de faire des propositions de faire avancer les choses, la référence à la loi de 2016, je crois qu'il est aussi importante, ce sont des références important alors pour conclure notre groupe les républicains suivra la position du président Philippe Bas, au nom de la commission des lois, je remercie, je vous remercie toutes et tous de votre attention. La parole est à monsieur Thani Mohamed dit. Monsieur le président, pour 6 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure mais chers collègues l'vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, la France peut Sanofi guérir de pouvoir compter sur une fonction publique de grande qualité, dénombrant plus de 5 millions de fonctionnaires parce qu'elles présentent une utilité réelle pour les fonctionnaires notamment Les Hauts fonctionnaires et leur employeur public la mobilité doit être encouragé à l'intérieur même de la fonction publique d'État, elle permet aux fonctionnaires de construire des trajectoires plus riche et d'acquérir une expertise sur des problématiques très diverses : entre le secteur public et le secteur privé, elle donne les outils pour appréhender de façon concrète les besoins des entreprises et des associations et participer ainsi efficacement à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques, enfin des échanges internationaux doivent occuper une place clé dans la formation continue Des aux fonctionnaires, car ils permettent de décentrer le regard et d'évaluer l'efficacité de nos techniques, administratives, la connaissance passer aux fonctionnaires des différents versants de notre fonction publique du fonctionnement des structures partenaires du secteur privé et du fonctionnement des administrations étrangères est un gage d'efficacité, néanmoins, si l'État et l'opinion publique attendent de leur aux fonctionnaires qu'ils soient opérationnels, ils attendent avant tout qu'il soit exemplaire, notre action publique et, par extension, les agents publics qui la composent doivent être au-dessus de tout soupçon, surtout au regard de la défiance actuelle de nos concitoyens inverse qui exercent une activité publique c'est dans ce contexte que notre assemblée examine la présente proposition de loi dans l'objectif vise à encadrer plus strictement la mobilité entre fonction publique, des fonctions privées aux fonctionnaires en renforçant les mécanismes de prévention des conflits d'intérêts liés à celle-ci, et notamment les compétences et les prérogatives de la commission de déontologie de la fonction publique, ce texte présente l'intérêt d'engager en séance publique, un débat sur la haute fonction publique et la prévention des conflits d'intérêts, ainsi que l'équilibre délicat à trouver entre nécessité d'encourager la mobilité et c'est indispensable, encadrement des conflits d'intérêts, néanmoins, la proposition de loi me me pose un réel problème de calendrier car elle survient soit trop tard, soit trop tôt et je m'en explique en effet la loi déontologie des fonctionnaires du 20 avril 2016 qui a permis d'élargir le périmètre de compétence de la commission de déontologie notamment sur toutes les questions relatives aux conflits d'intérêts et rendu obligatoire la saisine par l'agent public préalablement à l'exercice d'une activité extérieure n'est applicable que depuis un peu plus d'un an, elle n'a pour l'heure pas encore fait l'objet d'une évaluation pour mesurer l'efficacité des dispositifs qu'elle contient, il ne paraît dès lors prématuré de légiférer de nouveau sur ce sujet par ailleurs le groupe RDSE a présenté cette proposition de loi le 3 janvier dernier, soit moins d'un mois avant la remise du rapport de la mission de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts, menée par les députés, Fabien Matras et Olivier Marie-Madeleine dans un esprit de respect des travaux engagés par chacune des chambres, lieu était me semble-t-il préférable d'attendre et de laisser l'initiative parlementaire à ce qui avait engagé publiquement ce travail dès le mois d'août 2017 président ce n'est pas une raison pour que comme communion aussi dans ses excès, de sorte que, s'interrogeant sur l'opportunité d'autant que sur l'efficacité de ces dispositions, le groupe la République en marche, votera contre cette proposition de loi. Bien, la parole est à monsieur Pierre Yves Collombat pour 6 minutes pour le groupe communiste républicain et citoyen écologiste. C'est le président, merci. Monsieur le ministre, je vous salue, de nouveau, puisque nous sommes déjà vu ce matin. La la déontologie, c'est comme la médecine par les plantes. ça ne fait pas de mal. Mais qu'elle puisse guérir de vrais malades reste à prouver. Or les institutions. Les institutions de notre République sont sérieusement malades, comme le montrent les résultats électoraux de 2002 2017 véritable triomphe du dégagisme de l'absentéisme des votes blancs et nuls, les élus députés comme président de la République, l'ont été par défaut. Cette sécession civique renvoie pour une bonne part au sentiment que quelle que soit l'issue des consultations pour l'essentiel, la même politique continuera avec les mêmes résultats résultat qui marque la transformation progressive de la 5ème République en république oligarchique cogéré par la nébuleuse politique gravitant gravitant autour du président par les fondés de pouvoir des milieux d'affaires très grandes entreprises et par une nouvelle bureaucratie céleste.

donc constitué Ankara, selon l'expression, je n'invente rien d'Emmanuel Macron, lui-même. à ceux qui se protègent veille à son enrichissement. La fonction de l'État n'est plus de faire prévaloir à l'intérêt général, distincts des intérêts particuliers, mais d'assurer la pérennité du site du système, la concurrence libre et non faussée entre les acteurs, l'intérêt général résultant du bon fonctionnement du marché et non d'équilibre dont l'État serait le garant. Dans un tas d'agencement des pouvoirs le pantouflage mes allers-retours du public. Politique et administratif au privé, ont une fonction essentielle. Pas seulement, comme on le dit une gestion fluide des carrières de haut fonctionnaire, mais celle de l'Iran entre les membres de l'oligarchie, pas question donc d'interdire ces pratiques même pas dire limiter significativement. Les défenseurs du système sont très nombreuses, je constate encore première ligne de défense du pantouflage contre les irresponsables qui voudraient le réduire à la portion congrue premières lignes de défense donc noyer le poisson. Laisser croire qu'il est un phénomène qui reste marginal, selon l'expression même du récent rapport d'information de l'Assemblée nationale de février 2018,

Sauf qu'agrégé des inspecteurs généraux des Finances rouages rejoignant une grande banque des agents hospitaliers ouvre une pizzeria, les professeurs de philosophie de devenant Berger, ça n'a aucun sens. le privé n'est pas le nombre de fonctionnaires quittant le service public où y revenant mais que dire aux fonctionnaires ayant directement participé à l'élaboration des lois et des règlements, se retrouve en position de faire bénéficier leur nouvel employeur de leur connaissance intime des secrets des secrets de fabrication de leurs carnets d'adresses moyennant évidemment la multiplication plus que substantielle de leur salaire dans certains misent ministère et certains corps, celui des inspecteurs des finances, particulièrement le pantouflage, n'est pas une pratique marginale ainsi sur les 333 inspecteurs et inspecteurs généraux des Finances recensés par une enquête de 2017 plus de 55 pourcent travaillent ou ont travaillé dans le secteur privé, donc 34 pourcent dans le secteur bancaire, à un moment, leur parcours reviennent dans le secteur public, après avoir travaillé dans le privé, les allers-retours multiple étant près de 40 pourcent on fait un passage par un cabinet ministériel ou ont exercé un mandat politique, plus de la moitié des grands patrons français du CAC 40 sont polytechniciens ou énarques 2ème ligne de défense : réduire le problème du pantouflage extensif des grands corps à celui du conflit d'intérêt, à une simple question de déontologie, pas question de se préoccuper des effets corrosifs d'une telle pratique sur les fondements de notre démocratie, on se contente, on se concentrera donc sur les dispositifs techniques commission et entretient lui ontologie déclaration en tous genres, charte éthique censé prévenir les Lekodi conflit d'intérêt, quel est l'esprit de cette proposition de loi comme du rapport d'ailleurs de l'Assemblée nationale évoquée plus haut, je le cite : vos rapporteurs considèrent le dispositif légal actuel aboutit notamment grâce aux dernières évolutions donc circuler et après rien à voir 3ème ligne de défense un usage spécieux du conflit d'intérêt réduit au seul risque de favoritisme ainsi la seule contrainte qui s'impose, fonctionner à passer dans le privé et de ne pas faire bénéficier son nouvel employeur d'information donc ses concurrents disposerait pas un ancien directeur de BNP-Paribas, devenu gouverneur de la Banque de France devrait lui se déporter si l'institution doit traiter une question intéressante Paribas afin d'éviter tout traitement de faveur par rapport à ses concurrents, il ne vient pas à l'esprit que le risque de conflit d'intérêts pourrait se situer ailleurs entre les intérêts du système bancaire, opposé à tout ce qui pourrait ralentir son Business et ceux des citoyens avant tout préoccupés par la résilience du système bancaire aux crises spéculatives, le rôle joué par exemple c'était c'était évident par la Banque de France dans l'échec du projet de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires montre qu'il ne s'agit pas d'une question théorique non seulement la proposition de loi ignore ces questions essentielles non seulement dès le départ et s'en tient à quelques mesures déontologiques que l'on aurait pu soutenir visant à renforcer les dispositifs de contrôle existant, mais à l'arrivée, malgré la d'adoption de quelques de quelques amendements, il n'en reste plus grand chose, elle s'est auto-détruite en vol, difficile de s'y résoudre et de ne pas a réaffirmé qu'il faut en finir avec ces pratiques délétères. La parole est maintenant à monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE, il a 6 minutes. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois Madame le rapporteur, mes chers collègues, dans une interview parue le mois dernier, Marylise Lebranchu, revenant sur les circonstances qui l'avait conduit à abandonner une réforme des grands corps de l'État décrivez comment certains des membres au plus haut poste clé de l'État avait assiégé, ce sont ses mots, le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, afin de s'y opposer, l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen programme proclame pourtant que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, c'est le signe qu'une réforme de la haute fonction fonction publique ne pourra venir que du parlement et en particulier du Sénat, où l'on trouve encore quelques esprits libres étranger aux atermoiements d'un microcosme bureaucratique. Dans ces mêmes murs après le consensus qui s'est dessiné dans l'hémicycle au cours de l'examen de la loi sur la confiance dans l'action publique et dans un contexte très favorable après la publication du rapport d'information de nos collègues députés Matra Marlex nous éprouvons encore quelques résistances au changement, une fois la question posée frontalement l'identité des corps et plus tenace que d'autres partisane territoriale, la prévention des conflits d'intérêts et implique-t-elle de soumettre liés aux fonctionnaires des dispositions particulières et notamment d'encadrer davantage leur pratique de la mobilité, nous en sommes convaincus, comme vient de vous l'expliquer ma collègue Maryse Carrère il est encore possible de faire de belle carrière au service de l'État, à condition d'y entrer avec la conscience modeste d'intégrer un grand ensemble la question de la rémunération ne devrait pas être évitée pour autant, même si ce sujet reste souvent tabou en France, la mobilité des fonctionnaires est vital au cours de 40 ans de carrière, il faut l'encourager et la valoriser notre proposition de loi permet quelques améliorations nécessaires au dispositif créé par la loi, déontologie des fonctionnaires de 2016 destiné à prémunir Les aux fonctionnaires des suspicions qui pourrait naître du fait de leurs allers-retours entre le secteur public et secteur privé, voilà des mesures qui devrait contenter les partisans de la transparence, la clarification des règles relatives à la durée de la mise en disponibilité est également essentiel à nos yeux. Par le passé, la commission des lois, s'est souvent montré peu frileuse plus frileuse pardon que l'hémicycle pour légiférer sur ces questions, nous saluons à ce titre, le grand sens du devoir de notre collègue Josiane Costes qui bien que coauteur du texte la considérablement élagué en tant que rapporteur afin de parvenir à une version satisfaisante pour la majorité des membres de la commission des lois. Pour travailler ces auditions ont également permis de mettre en lumière 2 points importants : d'une part, la fusion avec la Haute autorité et de la commission déontologique qui devrait permettent de rendre les contrôles plus efficaces, nous avons donc déposé un amendement en ce sens à partir d'un amendement, déjà adopté par le Sénat, à l'initiative de Madame Di Falco, cela n'est d'ailleurs pas totalement contraire à un amendement adopté que vous aviez cosigné en tant que député, monsieur le ministre, qui prévoyait de donner compétence à la Haute autorité pour apprécier la déclaration d'intérêt des agents quand l'autorité hiérarchique n'était pas en mesure de le faire, l'autre point que je voudrais souligner la difficulté de soumettre la haute fonction publique à des règles particulières lorsque les nulle part défini le renvoie à la définition de périmètres des catégories A plus voir à plus plus à des décrets comme celui fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du seul gouvernement donne l'impression d'une haute fonction publique en autogestion, le trouvons laconisme de la loi concernant les règles mobilité à favoriser le maquis réglementaire actuel dont seuls les mieux informés finalement savent tirer profit pour conduire de longue carrière dans le secteur privé, sans abandonner la protection du statut de la fonction publique, n'y a-t-il pas une question déontologique, on cite souvent une phrase de l'ancien régime et la Révolution de Tocqueville pour s'opposer à la modification des règles imposées aux grands corps de l'État depuis 1789 je cite la constitution administrative est rester debout dans les cendres des constitutions politiques. Il en est ainsi suggérer que face à la volatilité des opinions politiques des Français, l'administration, seule la continuité de l'État. Cet l'esprit de cet ouvrage où il est écrit par ailleurs les phrases suivantes qui d'une certaine manière, éclairent les circonstances particulières de nos débats, je cite : les fonctionnaires administratifs presque tous bourgeois forment déjà une classe qui a son esprit particulier, ses traditions, ses vertus son honneur, son orgueil propre, c'est l'aristocratie de la société nouvelle qui a déjà formé et vivante, elle attend seulement que la révolution vidé sa place, ce qui caractérise déjà l'administration enfance c'est la haine violente que lui inspire indistinctement tous nos bourgeois qui veulent s'occuper des affaires publiques, en dehors d'elle, a un mot Edmonton point que les citoyens s'ingère d'une manière quelconque dans l'examen de leurs propres affaires, elle préfère la stérilité à la concurrence, fin de citation chaque collègue nous espérons donc que le vote de cet après-midi ne sera pas stérile mais cohérent avec les positions précédentes prises par notre hémicycle dont le monde du 21 février dernier un collectif de haut fonctionnaire a publié une tribune intitulée la haute administration, le véritable parti présidentiel Tribune faite par un collectif de hauts fonctionnaires qui estime que le macronisme, entre guillemets, se distingue par à confusion entre une partie de la haute administration et la politique du gouvernement, la haute administration et donc déjà sous les feux de la rampe et il est de notre responsabilité de ne pas la laisser en proie à une sorte de vindicte populaire ne pas légiférer, aujourd'hui, c'est se condamner à devoir le faire dans quelques temps, sous la pression et nous savons tous que sous la pression, la passion pourrait prendre le pas sur une réforme objectif des choses objectivité rappelée par le président de la commission des lois à l'occasion des différentes réunions ne pas légiférer aujourd'hui comme nous le proposons, c'est un manque de discernement, la presse est déjà attentive au sujet que nous abordons quant à l'argument tiré du respect de l'Assemblée nationale, je ne ferais pas partie de ceux qui font des courbettes à l'Assemblée nationale le bicamérisme français ne passe pas par la soumission des travaux d'une assemblée à une autre, mais bien par le respect de l'indépendance de chacune d'entre elles. y a la discussion générale est Close, nous passons à la discussion du texte de la Commission et avant l'article 1er il y a l'amendement numéro 12. Présenté par Madame Maryse Carrère. Vous avez la parole. Merci monsieur le président. Alors, mes chers collègues, lors de ses auditions, notre rapporteur, a constaté la difficulté de soumettre Les aux fonctionnaires à des exigences particulières en matière de lutte contre les conflits d'intérêts alors ce en raison de l'absence de définition légale, il existe une appellation officieuse, la catégorie A Plus qui est actuellement utilisé pour désigner les fonctionnaires de catégorie A, bénéficiant de traitements supérieur à la moyenne de la catégorie en raison de leur fonction supérieur dans la hiérarchie administrative d'autres interlocuteurs de la rapporteure ont également évoqué l'appellation j'ai 16 pour les 16 degrés encore, mais cette appellation si semble davantage reposer sur des critères honorifique sur un tout autre sujet était récemment évoqué la revendication des gardiens de prison d'être considérés comme des agents de catégorie B en constate donc bien qu'à raison du gel du poignet indices et des diverses qu'à Sion qui en découlent, la fin des frontières des catégories classiques sont remises en cause dans ces conditions et dans le cadre d'un travail de réflexion globale sur la rémunération des agents publics, la création d'une d'une nouvelle catégorie supérieure à la catégorie A pourrait être envisagée, rassemblant les corps destiné à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, il s'agit d'une revendication du haut fonctionnaire qui pourrait également être utile pour renforcer la prévention des conflits d'intérêts, les concernant, c'est pourquoi un rapport du gouvernement pourrait nous éclairer en la matière, c'est ce que nous demandons avec cet amendement. Merci l'avis de la commission Madame. Effectivement, les auditions que j'ai menée dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi m'ont permis de constater et de regretter qu'il n'existait aujourd'hui, pas de définition légale de la haute fonction publique cette absence de définition légale conduit selon les interlocuteurs que j'ai entendu à des évaluations différentes du nombre de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire de ceux appartenant à la catégorie non officielle à plus leur nombre serait compris entre 12000 et 34000 personnes, sans compter les maîtres de conférences, de même je n'ai pas pu obtenir de données précises sur la mobilité des fonctionnaires vers le secteur privé, il serait donc intéressant que le gouvernement se dote de notices plus étoffé la commission des lois, une position en sait ancienne et constante sur les demandes de rapport, elle n'est pas favorable, nombre d'entre eux Nombre de ces rapports ne sont jamais remis, en dépit des demandes du Parlement, en outre, rien n'empêche des assemblées au titre de leur mission de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, de créer une mission d'information où une commission d'enquête sur ce sujet, c'est donc un avis défavorable de la commission des lois. Oui, Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, c'est un avis défavorable de la même manière, pour 2 raisons : la première, c'est qu'il n'existe pas définition statutaire, la catégorie la plus c'est une appellation qui concerne essentiellement les corps représenté, ce que vous avez évoqué tout à l'heure le j'essaie, c'est-à-dire l'association des syndicats ou d'associations représentant Les Hauts fonctionnaires ou les corps, recrutant à la sortie de l'ENA ou de Polytechnique, donc c'est la la première raison qui nous amène à nous opposer à la production de ce rapport, l'absence de bas statutaire, la 2ème tient à l'objet de la proposition de loi que vous nous vous nous proposez vous défendez des obligations déontologiques spécifiques aux emplois supérieurs la ministre à Sion, à savoir depuis 2013, des employes à la décision du gouvernement et, depuis la loi de 2016 les employes dans le niveau hiérarchique et la nature des fonctions le justifie ces emplois sont tous soumis à des obligations déclaratives, déclarations d'intérêt de situation patrimoniale, voire pour certains employes des mandats de gestion sans que leur appartenance ou non à ce qu'on appelle la catégorie la plus mais une incidence sur la situation, l'entrée par le prisme à plus ne suffit pas, finalement atteint l'objectif qui est le vôtre, matière déontologie pour les postes de fonctionnaires. Merci monsieur le ministre, il y a-t-il une explication de vote oui.

Qui s'abstient, cet amendement est rejeté. à l'article 1er. L'amendement 17 rectifié présenté par Monsieur Collombat. Il s'agit de réintroduire donc un un article qui était dans la proposition de de loi initial et et dont l'objet est de s'assurer une obligation donc que Les avantages pécuniaires que

avant de passer dans le privé, alors on va me faire on me fera bien sûr remarqué parce qu'on a déjà fait mais la plupart des gens sont en situation de disponibilité, donc il ne quitte pas la fonction, la fonction publique, sauf que ça peut durer sinon ad vitam eternam, du moins un temps intéressant certains et je voudrais quand même aussi faire remarquer. Que ces gens qui se présentent à des concours de recrutement. Prestigieux. Et qui s'en vont au bout de 2 ans ou 3 ans, ils prennent la place d'autres. Qui n'ont pas leur chance. Donc je trouve ça profondément illégitime. Un engagement en général ne sont pas très, très long, ses engagements. Quand on a pris un engagement, on le tient. L'avis de la commission Madame. Merci Monsieur le Président, le présent amendement soulève la question du remboursement des frais de scolarité pour les fonctionnaires demandant une mise en disponibilité avant le respect de leur engagement minimal au service de l'État, il semble opérer une confusion entre mise en disponibilité d'émission de fonctionnaires dans le cadre d'une mise en disponibilité le fonctionnaire 17 détiennent toujours un lien avec l'administration, aucune disposition de interdit aujourd'hui un jeune fonctionnaire de partir indisponibilité, quelle qu'en soit d'ailleurs le motif, on peut le regretter mais gardant à l'esprit qu'une mise en disponibilité limitée dans le temps avec des durées variables selon les cas. Dans le cas d'une démission et dans le cas où celle-ci interviendrait avant que soit respectée la durée minimale de leur engagement de service donc de servir dans la fonction publique, les fonctionnaires sont tenus de rembourser la pantoufle mais suivant les corps, la période de scolarité n'est pas toujours pris en compte cette obligation est donc prévu mais relèvent du domaine réglementaire, c'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable de la commission des lois. Merci la vidéo gouvernement Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, c'est un avis défavorable, pour des raisons identiques Assélé évoqués par Madame le rapporteur et d'autres raisons que j'ai présenté d'abord pour dire cet amendement selon nos ferait obstacle à la mobilité des carrières entre l'emploi public et l'emploi privé puisqu'il priverait tout fonctionnaire de la possibilité d'exercer une mobilité vers le secteur privé tant que son engagement de servir n'est pas satisfait, or cet engagement pour être satisfait, nonobstant une mobilité dans le secteur privé, c'est ce que l'on constate dans la plupart des cas, il faut aussi souligner que le décret du 9 mai 2017 relatif à la position disponible de disponibilité des fonctionnaires de l'État souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, vrai que lorsque l'engagement de servir n'a pas été intégralement réalisé la durée de la disponibilité pour convenance personnelle pour exercer des activités, donc dans le secteur privé est fixée à 3 ans renouvelable seulement une fois pour une durée d'un nom et le bénéfice d'nouvelle disponibilité de ce type est subordonnée à l'accomplissement de l'intégralité de la période, donc je m'en servir et enfin sur le plan rédactionnel, la notion de frais de scolarité, à la différence de celle de coups de scolarité n'est applicable qu'aux écoles de service public qui accueille également des élèves non fonctionnaires au-delà de ces frais et dans le cas des écoles n'ayant que des les fonctionnaires, il n'y a pas de frais de scolarité.

Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, donc il n'y a pas lieu de voter sur l'article qui était supprimée après l'article 1. L'amendement de rectifier Maryse Carrère oui, vous avez la parole. Merci, mes chers collègues, cet amendement avait déjà été adoptée par notre haute assemblée lors de l'examen de la loi sur la confiance dans l'action publique en juillet dernier à l'époque, la commission des lois, l'avait gratifié d'un avis favorable, chose exceptionnelle pour une demande de rapport, cette disposition n'avait pas été vaine, puisqu'elle avait en quelque sorte, conduit les députés, les députés Fabien Matras et Olivier Marlex à ouvrir une mission d'information qui a donné les résultats que l'on sait donc comprenant donc pas l'évolution de la commission sur ce point-là, de même que sur les amendements de 13 14 et 15 qui sont en réalité les amendements de Monsieur Jacques Genest, que le Sénat avait adopté cet été également, cette fois-ci, avec l'assentiment de la commission merci. Bien dans la discussion commune Monsieur Collombat le 24 actif. Il est défendu, c'est le même, il y a bon pas complètement Madame Coste, au nom de la commission. Merci Monsieur le Président, pour les mêmes raison de principe tenant à l'inanité des demandes de rapport au gouvernement qui sont rarement suivies d'effet et au pouvoir d'investigation des assemblées qui leur appartiennent, d'utiliser pour se venger pour leur propres analyses, c'est un avis défavorable de la commission des lois. monsieur le ministre, votre avis. les mesures relatives au remboursement des frais de scolarité ont été prises en 2014 en 2015 pour ce qui concerne l'ENA et techniques pour 2015 et l'économie normale supérieure en 2014 aussi, le 6 juin donc, les choses sont d'ores et déjà arrêté encadré. Bien on va procéder au vote sur chaque amendement, même si l'allié commun parce qu'ils sont presque identiques n'est pas identique formellement donc le de rectifier, qui est pour.

En fait, qui ne reprendra vie que si ces amendements sont adoptés. Amendement numéro 3 Maris Carrère, vous avez la parole. Merci, cet amendement vise à clarifier la rédaction du 3 de l'article 25 optimiste de la loi du 13 juillet 1983 qui décrit la procédure de saisine de la commission de déontologie 6 cas contraire les effort aux fonctionnaires soumis à déclaration de Patrimoine auprès de la HATVP de faire l'objet d'un contrôle de déontologie, renforcée par la commission de déontologie actuellement la saisine et confié concurremment aux fonctionnaires ou à son autorité hiérarchique, puis, en dernier recours par voie d'autosaisine au président de la commission de déontologie lui-même la multiplication des saisines 10 possibles est de nature à introduire de la confusion à dédouaner chaque partie de la responsabilité de saisir la commission de déontologie, pourtant obligatoire afin qu'elle soit mieux appliquée dans la pratique et de clarifier les dispositions existantes, il est donc proposé de faire porter la responsabilité de saisir la commission de déontologie à l'autorité hiérarchique uniquement notre il est proposé d'introduire une gradation Anne, ajoutant que les départs aux fonctionnaires, déjà soumis à obligation de transmission de déclaration de Patrimoine à la Haute autorité vers le secteur privé, font l'objet d'une auto-saisine par la commission de déontologie, il s'agit d'introduire de la subtilité, dans le dispositif, créé par la loi de déontologie afin que les contrôles portent prioritairement sur les personnes dans les fonctions sur les puces invincible, actuellement, en effet, la Commission des déontologie contrôle indistinctement les départs des agents publics, quelle que soit leur niveau de responsabilité pourtant, comme le disait DES récemment le député Olivier Marlex lors d'une interview délibérément Les Hauts fonctionnaires ont été mis de côté, or, c'est au tour 2 que se concentrent les conflits d'intérêts les plus dangereux, merci. Peut-être rester au micro pour votre amendement de repli numéro 4. Donc c'est votre collègue Monsieur Artano. Et qui vont-elles président c'est le l'amendement qui est identique à celui que risques carrière vient de présenter à la seule différence, c'est qu'il ne prévoit pas une c'est une auto-saisine obligatoire de la commission déontologie pour les fonctionnaires. Toujours dans la discussion commune le 18 rectifier Monsieur Collombat. il y a un triple objectif cet cet amendement, c'est proposer que la saisie préalable de la Commission en cas de décision définitive cessation définitive ou temporaire de ses fonctions par un fonctionnaire ne soit applicable qu'au fonctionnaires occupant un emploi public nécessitant une déclaration à la à la HATVP deuxièmement et tendre de 3 à 5 ans la durée contrôlée par la commission déontologie qui permet de mieux apprécier la la compatibilité des fonctions s'assurer, c'est la 3ème point s'assurer qu'en cas de non saisi la commission par le fonctionnaire, le président de la commission puissent le faire, s'agissant de certains employes sensibles dans la haute fonction publique, là encore, il s'agit pour pour moi pour nous d'un établir une distinction entre les fonctionnaires qui ont vraiment eu des responsabilités ou qui auront des responsabilités dans la fabrication de la loi et son application dans l'élaboration de sa jurisprudence et puis les autres, et dire que c'est pas la même chose, encore une fois que j'ai tout à l'heure un agent hospitalier ouvre une pizzeria, c'est pas le même problème que

Merci là l'avis de la Commission sur ces 3 amendements Madame Coste. Merci Monsieur le Président, bon pour la la les amendements 3 et 4 on demande l'avis du gouvernement pour l'amendement 18 main cet amendement propose 3 modifications majeures concernant les missions et les prérogatives de la commission déontologie de la fonction publique toute pose des difficultés en 1er lieu pourquoi restreindre le Champ de la saisine de la commission à la cessation temporaire ou définitive des fonctions des seuls fonctionnaires soumis à des des obligations déclaratives, alors qu'elle est aujourd'hui compétente pour l'ensemble des fonctionnaires les confiner intérêt ne concerne pas seulement Les aux fonctionnaires mais bien l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur catégorie leur corps et leur grade en 2ème lieu l'extension de 3 à 5 ans de la durée de contrôle assuré par la Commission déontologie peut sembler séduisante, mais il faudra prendre en compte les moyens humains dont dispose la Commission déontologie en fait c'est un secrétariat de 5 personnes pour assumer une telle extension cela rallonge aurait nécessairement les doubler les délais d'examen qui sont déjà critiqués pour leur longueur en 3ème lieu concernant la saisine de la commission par son président, là encore qu'une telle disposition soit opérante, encore faut-il que le président soit informé ou dispose des moyennes d'être informé d'un changement d'affectation de fonctionnaires, l'actuel président de la Commission, monsieur Roland m'a indiqué ne pas pouvoir être en mesure d'appliquer une telle saisine donc s'étonne d'une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable de la commission des lois. Merci madame, monsieur le ministre, votre avis sur ces 3 amendements. Merci Monsieur le Président, sur les Allemands non numéro 3 et numéro 4 présenté par Madame Carrère et monsieur Arnaud c'est une demande de retrait ou à défaut défavorable mais une demande de retrait pour les raisons suivantes l'état du droit oblige déjà tout fonctionnaire qui souhaitent partir, que ce soit temporaire ou définitif dans le secteur privé à saisir préalablement son administration et c'est cette même administration doit ensuite obligatoirement saisir pour avis la commission déontologique, il est possible à l'agence saisir directement la Commission mais cela représente dans la réalité, moins de 10 pourcent des saisines et dans cette hypothèse, la commission n'avertit systématiquement l'administration afin de recueillir notamment son appréciation sur le projet professionnel de l'agent sur le B de votre amendement madame présenté par Madame Carrère, les agents soumis à l'obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale au titre du de l'article 25, inquiète de la loi du 13 juillet 1983 entre déjà dans le Champ de la saisine obligatoire, la commission d'anthologie et donc l'état du droit satisfait l'amendement que vous avez présenté, et c'est la raison pour laquelle, pour les amendements 3 et 4, je répète, c'est une demande de retrait aussi ils étaient maintenus, un avis défavorable pour l'amendement numéro 18 c'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par Madame le rapporteur, j'ajoute simplement que pour le gouvernement, le 2ème point d'amendement qui consiste à étendent la durée sur laquelle porte le contrôle de la commission déontologie nous sommes de nature à faire obstacle à la fluidité des parcours professionnel exigeant public quelque que soit leur catégorie alors que nous considérons que cette fini es peut-être un élément d'attractivité de la fonction publique. Alors il y a une demande de retrait de la part du gouvernement, des amendements 3 et 4 je me tourne vers leurs auteurs. Pour les maintenait.

alors sur le 4, la Commission avait demandé l'avis du gouvernement qui a dit : retrait et n'est pas retiré et que donc il a dit défavorable, donc la commission avec cet avis du gouvernement, nous dit quoi maintenant. Avis défavorable et donc avec 2 avis défavorables je le soumet au vote qui est pour. Qui est contre. On va compter. Qui est pour. Qui est contre.

Après l'article de nous sommes à l'amendement numéro 5. Madame Carrère monsieur Artano monsieur Artano le défend. Merci monsieur le président, cet amendement vise à réintroduire une disposition présents dans le texte initial et qui visait à ce qu'une procédure disciplinaire soit engagée obligatoirement en cas de non respect de la vie d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, la commission déontologie les rapporteurs Matra Marlex on aboutit aux mêmes conclusions que nous si les administrations ne s'assure pas que les avis avec réserve ou d'incompatibilité sont effectivement respecté alors ces avis ne seront effectivement que des gadgets, notre objectif est et plus précisément la des gadgets des dispositifs prévus en 2016 et cela passe par un meilleur suivi des avis de la commission, ouverture d'une procédure disciplinaire en cas de non, respect mais également la publication des avis, ce qui a été justement proposé par notre rapporteur, ainsi que le suivi des fonctionnaires en situation de pantouflage permis par votre amendement 9 sans les moyens de renforcer le texte de 2016. Madame Coste pour la Commission va être ravi. Merci Monsieur le Président, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un fonctionnaire qui n'aurait pas respecté les avis de la commission déontologie de la fonction publique rendue à son encontre, il serait ainsi mis fin au pouvoir d'appréciation de l'autorité hiérarchique à la matière mais pourquoi dans ce cas seulement, et pas pour d'autres comportements fautifs, la Commission considère que l'administration doit conserver son pouvoir d'appréciation en fonction de la nature et de la gravité de la faute commise la commission donc propose un avis défavorable. La vision gouvernement Monsieur le Ministre. C'est le même avis Monsieur Président défavorable car la disposition proposée par cet amendement conduirait à placer le chef de service dans un agent de respecteraient pas l'avis de la commission en Suisse sont de compétence qui pour ouvrir une procédure disciplinaire, avec un effet déresponsabilisation pour lui-même et l'impossibilité d'apprécier l'intensité du manquement constaté au cas par cas, comme vient de le rappeler Madame la rapporteur. Il y a-t-il une explication de vote Monsieur Bigot.

la déontologie, c'est quelque chose qui est interne au corps, donc c'est le corps qui doit savoir s'il renvoie quelqu'un en conseil de discipline, si nous considérons qu'il faut qu'il y a un regard extérieur, il faut trouver d'autres dispositions ce que des non-respect de règles déontologiques sont faites par exemple par des professions libérales soumises à un ordre l'ordre peut se saisir, mais le procureur de la République peut également saisir

Non, contre cet amendement, Qui a été supprimée, mais qui peut revivre un de ces amendements est adopté le 19 rectifier Monsieur Colomba, vous avez la parole. De de modifications par rapport à l'ordre actuel à l'amendement donc il étant le recrue qui étant le recrutement donc des magistrats qui interviennent dans la dans la commission au-delà du Conseil d'État et de la Cour des comptes, donc c'est ce que nous proposons, c'est que les magistrats moins moins élevés que ce qui existe actuellement, puisse participer donc constitue le le collège de la de la Commission et, ensuite, s'agissant des personnalités qualifiées qui actuellement sont personnes, de lancer une appartiennent donc à des entreprises privées a plutôt leur préférer des personnalités qu'on connus par leurs travaux et leur expérience, les questions de conflit d'intérêts ou de prévention de la corruption, parce que c'est, c'est un principe c'est ça quand même

bien de l'avis de la commission madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président pour éviter l'entre-soi dénoncée par notre collègue le conseiller d'État serait remplacé par un magistrat de l'ordre administratif le conseiller maître à la Cour des comptes, par un magistrat financier et des personnalités qualifiées choisies en fonction de leurs travaux sur les conflits d'intérêts. Les auditions que j'ai menée pour l'examen de cette proposition de loi n'ont nullement soulevé les difficultés particulières relatives à la composition de la commission déontologie de la fonction publique, en outre, les critères de choix des personnalités qualifiées, me paraissent très vague, on peut imaginer que ce soit des universitaires qui seraient en priorité choisie, or si aujourd'hui une personnalité qualifiée sur les trois et choisi pour avoir des exercer des fonctions dans le secteur privé, c'est justement pour avoir une expertise de la part de quelqu'un qui connaît le secteur privé, de l'Intérieur, c'est un aspect essentiel pour apprécier la compatibilité des fonctions entre secteur public et secteur privé, en fait, nous avons adopté l'amendement numéro 16 cet amendement est donc contraire à celui-ci puisque la maman numéro 16 reprend la commission actuelle de la Commission déontologie de la fonction publique, la commission des lois émet donc un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, à l'exception de l'argument utilisé par Madame le rapporteur sur le fait que la Commission et adoptées, l'amendement grossesse bien sûr ce sont les mêmes raisons qui nous amène à donner un avis défavorable. Très bien, il y a-t-il une explication de vote Monsieur Collombat. J'ai un peu, un peu du mal à comprendre les explications ou l'absence d'explication qui m'a été donné, et dire que qu'est-ce que ça peut avoir de de scandaleux qu'on élargisse le Champ de de recrutement donc des magistrats qui font, qui composent la commission

le problème c'est pas de savoir si ça serait intéressant pour les entreprises, encore une fois de faire telle ou telle recrutement c'est c'est d'avoir une

Qui est contre qui s'abstient, il est rejeté, article 4. Maryse Carrère ou Monsieur Artano vous avez la parole. Merci Monsieur le président, c'est un moment est important, il permet de s'assurer de l'effectivité de la prévention des conflits d'intérêts, au moment de la réintégration d'un fonctionnaire, après une période de pantouflage sur une période de 3 ans, et non uniquement au moment de la réintégration, il permet en quelque sorte d'aménager un sas de réintégration sur lequel un fonctionnaire pourrait demander à être réintégrée dans un service conforme puis changer de service, quelques mois après et se retrouver en situation de conflit d'intérêts, cette disposition ne relève pas davantage du gadget. L'avis de la commission, même la rapporteure. et son retour dans le secteur public changerait d'affectation dans le secteur public, moins de 3 ans après son retour dans l'administration, cet amendement permettrait de contrôler des voeux d'éventuels abus de fonctionnaires qui, pour échapper au contrôle de la commission déontologie de la fonction publique occuperait Tom 1er poste avec un habit de compatibilité de la commission avant d'effectuer une mobilité dans un délai assez court pour occuper un nouveau poste qui pourrait soulever des questions de compatibilité donc sur sur cet amendement, la Commission s'en remet à la sagesse du Sénat. y a monsieur le ministre, votre avis. Merci Monsieur le Président, le gouvernement considère que l'objectif poursuivi par les auteurs est satisfait, notamment par les dispositifs créé par la loi du 20 avril 2016, telle que la déclaration d'intérêt pour prévenir les conflits d'intérêts avant la nomination sur certains emplois. Vous craignez, comme l'a dit Madame le rapporteur, que le retour dans la fonction publique se fasse sur un emploi faisant l'objet d'un avis favorable et qu'ensuite les nominations sur un emploi plus sensible et qui aurait été peut-être plus difficile d'accès, ces emplois plus sensibles qui ont été listés par le décret du 28 décembre 2016 font l'objet d'un examen avant la nomination, donc c'est la raison pour laquelle nous considérons votre objectif est satisfait et ça n'a l'idée favorable à défaut de rentrer. Eh bien, il y a cette demande de retrait. Dites le plus fort, j'entends pas donc sagesse de la part de la Commission défavorables de la part du gouvernement qui est pour.

qui est pour. Qui s'abstient, il est adopté. Donc 3 amendements en discussion commune. Le vent a rectifié Monsieur Colomba, vous avez la parole. Bien Bien cet amendement donc vise à interdire à certains fonctionnaires précisément désignés d'Europe pour revenir au pouvoir revenir exercer un emploi dans la fonction publique qui recouvre la même le secteur l'équité que celui qu'il occupait dans le privé en limitant très strictement

Merci Monsieur le Président, c'est un moment vise à préciser la liste aux fonctionnaires devant faire l'objet d'un contrôle de la commission de déontologie au moment de leur réintégration, plutôt que de laisser cette tâche au Conseil d'État, ce qui aurait pour conséquence de retarder l'entrée en application, nous avons bien conscience qu'il n'est pas très satisfaisant de légiférer en établissement des listes à la Prévert mais cette façon de faire, a déjà été utilisée lors de la loi Sapin II notamment cette rédaction a donc le mérite de la clarté et d'une grande exhaustivité même que la solution alternative proposée à l'amendement suivant. Merci et poursuit avec la demande mon numéro 10 Madame Carrère. Eh oui, il s'agit d'un amendement de repli, Yves Izard un périmètre plus restreint sur la base du décret en Conseil d'État a pris en application de l'article 25 à une caisse de la loi de de 1983 après sa modification par la loi de déontologie. nom numéro 1 de cet amendement pose un principe général selon lequel haut fonctionnaire revenant du secteur privé ne pourraient pas occuper de postes au sein du secteur public, dans le même domaine d'activité que celui qu'il occupait dans le secteur privé, je rappelle à notre collègue que la commission des lois à mon initiative a étendu le contrôle de la commission déontologie de la fonction publique, au retour d'un fonctionnaire dans le secteur public, après avoir occupé des fonctions dans le secteur privé, il reviendra dans ce dans dans ce cas à la Commission d'apprécier la compatibilité entre les fonctions passées dans le secteur privé et celle que souhaiterait exercer le fonctionnaire à son retour dans le secteur public il ne semble donc pas pertinent de prévoir une interdiction générale de principe, ce n'est pas, ce n'est pas le secteur d'activité qui doit primer, mais l'émission effectivement exercées par un fonctionnaire lors de son retour dans le public,

amendement numéro 7 c'est un avis favorable de la commission des lois. Et donc, comme l'amendement numéro 7 a reçu un avis favorable donc ces demandes de retrait ou pour l'amendement numéro 10 ou 11 il satisfait par l'amendement numéro 7. C'est bien l'avis du gouvernement Monsieur le midi sur ces amendements. Merci Monsieur le Président, sur l'amendement numéro 20 l'avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le rapporteur sur les amendements suivant le numéro 6 c'est une considérant que le décret du 28 décembre 2016, qui fixe la liste des des emplois donnant lieu obligatoirement une déclaration d'intérêts est un dispositif suffisant pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêt pour leurs futurs occupants titulaire et donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. nous allons passer au vote sur chacun de ces amendements, l'amendement va rectifier 2 avis défavorables qui est pour. J'ai contre. Qui s'abstient, il est rejeté ensuite l'amendement numéro 7, un avis favorable de la commission et un avis défavorable. Sa demande de retrait de la part du gouvernement, il n'est pas retiré, donc avis défavorable, gouvernements, qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient, il était adopté, et celui-là est satisfait donc tombe, c'est un amendement de repli, bon nous passons maintenant, nous allons d'ailleurs passer on va vous votez l'article IV dans son ensemble qui est pour.

je comprends parfaitement, madame la rapporteure votre volonté qu'il y avait un un contrôle au moment du retour mais il peut paraître dangereuse, le contrôle d'abord, il doit se faire par les gens qui vont nommer le haut fonctionnaire dans le poste, ou le fonctionnaire dans le poste qu'il souhaiterait intégrer c'est à d'abord de vérifier la compatibilité et le fait de d'obliger de saisir obligatoirement la commission de déontologie peut poser un problème ultérieurement admettez que néanmoins 7 personnes soient poursuivis par un procureur de la République pour les infractions prévues par le code pénal et visé dans votre article. Ce fonctionnaire pourra dire mais j'ai interrogé la commission déontologie qui m'a donné un avis qui a donné un avis et qui considère qu'il n'y a pas tremblé donc ça ouvrira un débat après tout, un de plus, mais cela prouve bien que, en allant sur ce texte, un peu trop vite nous ne mesurons pas complètement les conséquences donc je suis favorable à ce qu'il y ait ce type de contrôle mais faisons très attention, c'est plutôt à l'administration qui renomme qui doit vérifier plutôt que de dire on saisit une commission d'déontologie, je pense que c'est toute l'erreur du texte. Qui est pour l'article IV.

Il s'agit simplement de de rendre publics tous les avis, donc de la commission de déontologie. Merci pour cette sobriété madame Maresca Scraire Monsieur Artano sur l'amendement numéro 8 ah pardon, non, non, ils sont pas discussion commune, on va les aborder un parrain Madame Coste votre avis. L'objectif de cet amendement est déjà satisfait par la guerre, la rédaction de l'article 4 bis de la proposition de loi en outre son Champ d'application est moins large puisqu'il ne concernerait que certains avis rendu par la commission déontologie de la fonction publique, alors alors que le texte adopté par la commission les visent tous, donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci monsieur le président, l'avis du gouvernement est défavorable car nous considérons que cet amendement ne respectent pas l'état de droit en vigueur concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel et qui l'emporterait également du fait d'une impression de rédaction risque d'incompétence négative du législateur et nous rappelons que sur le fond, il faut rappeler que la commission rend déjà publique un rapport annuel, dans lequel elle analyse en respectant le secret de la vie privée des agents concernés les avis qui sont rendus le Net et me commande de dire que de manière générale, le gouvernement ne partage pas l'article 4 de la rédaction, qui a été arrêté à l'occasion de l'examen en commission puisque nous considérons là aussi qu'il y a un risque en matière de respect de la vie privée d'un certain nombre de ces dispositions et que nous, nous considérons que la rédaction ne correspond pas à l'exposé des motifs de l'amendement, puisque l'exposé des motifs, vise à ce que les administrations soient informés des décisions rendues par la Commission, ce qui est déjà le cas pour tous les agents qui saisissent la commission d'déontologie et non pas une publication intégrale des avis. Merci, y a-t-il une demande explication de vote. Bon, je ne vois pas, nous allons passer au vote, avec demande de retrait ou autres iraient pas donc 2 avis défavorables. Qui est contre Qui est contre qui s'abstient, il est rejeté, on passe à l'amendement numéro 8. Carrère. Où il y a en l'état actuel, l'article 4 bis laisse à la commission de déontologie de fixer elle-même les conditions de publication des avis de réserve d'incompatibilité afin d'éviter les délais d'un ancrer en vigueur, il est proposé de préciser la rédaction et de prévoir que les avis anonymiser son ne soit publié, selon les règles d'anomie n'immunisation passa dire déjà prévue par le code des relations entre le public et l'administration. L'avis de la commission Madame Coste. C'est un avis favorable. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le président, nous considérons que dans la mesure où l'anonymisation ne concernerait que le patronyme de l'agent concerné ainsi que le cas échéant, le nombre d'entreprises qui souhaitent procéder à son recrutement et que la publication descriptif exhaustif et près exhaustif pardon et précis des fonctions exercées par l'agent est de nature à permettre aisément son identification, tout cela est de nature à méconnaître le droit au respect de la vie privée énoncés à l'article 8 de la CEDH protégé par la Constitution, donc en encourir avec le l'appréciation très très réservé du gouvernement sur l'article 4 bis, la vie ne peut-être que défavorable. Mais nous allons passer au vote qui est pour cet amendement, il y a un avis favorable, la Commission à l'avis défavorable du gouvernement. Qui s'abstient, Qui s'abstient, il est adopté, nous passons au vote de l'article 4 bis dans son ensemble qui est pour. Qui est contre elle est adoptée. Je mets au voilà 5 qui est pour. Qui est contre, il était adoptée après l'article 5 en discussion commune un amendements et sous-amendements. Mais, mais c'est pas écrit. Donc 2 sous-amendements. Le 16 rectifier bis Madame Carrère,

Cet amendement vise à transférer les compétences de la commission de déontologie à une commission spécialisée de la HATVP ce, spécialement créé sur la base de la main demain de Madame Di Folco que le Sénat a déjà adopté, il est enrichi de la publicité des avis de la commission du contrôle du personnel des et des API de la faculté pour cette commission d'assurer une contrôle à la réintégration des agents, ce qui est également conforme aux préconisations du rapport Matra Malak cette fusion est justifiée par les compétences concurrentes qu'exerce aujourd'hui la HATVP, la commission de déontologie a matière de lutte contre et confident intégrer et VP étant chargé du contrôle des déclarations de Patrimoine, certains hauts fonctionnaires, cette fusion et bien sûr perfectible, la composition de la commission spécialisée pourrait être revu si c'est trop position de loi poursuivait son chemin législatif, il s'agissait pour nous de parvenir à une compromis Haffen établir une base de discussion entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Merci la les sous-amendements, ça peut être vous, monsieur, puisque vous êtes signataire des sous-amendements. Merci monsieur Merci monsieur le président. Donc le sous-amendement numéro 28 est un amendement de précision qui vise à introduire un sas de 3 ans après la réintégration d'un haut fonctionnaire, après l'intégration de la commission spécialisée par la HATVP, le sous-amendement numéro 29 vise également à préciser le dispositif de fusion définissant le périmètre aux fonctionnaires concernés par le contrôle au moment de la réintégration comme l'amendement précédent concernant la commission déontologie. L'avis de la commission Madame Coste sur ces amendements et sous-amendements. Donc ces 2 sous-amendements n'ont pas été examinés par la commission des lois, en raison de leur dépôt tardif, l'amendement numéro 6 ayant état ayant été adopté avec l'avis de sagesse de la commission, je donnerai tout du personnel, un avis favorable au sous-amendement numéro 28 qui le reprend par cohérence l'amendement numéro 7 ayant été également adopté avec l'avis favorable de la commission, je donne donc un avis favorable au sous-amendement numéro 29 qui le reprend toujours par cohérence.

Merci Monsieur le Président, sur l'amendement d'abord et, par conséquent, cela sous-amendements, sur l'amendement la proposition suscite de nombreuses réserves au moins 2 d'abord, cet amendement nous permet, pardon, de souligner qu'il existe une réelle différence. Entre la commission déontologique qui allie l'expertise globale sur la question déontologie de l'ensemble des agents publics et l'examen des situations individuelles de ceux d'entre eux qui part dans le secteur privé concurrentiel et la Haute autorité qui contrôle l'exemplarité, notamment l'absence de conflits d'intérêts et une intégrité financière de ce agents publics ou non occupant des emplois en proximité forte avec l'autorité politique, la 2ème réserve qui en fait que pour celle de leurs compétences, qui appelle une coordination, la Commission et la autorité ont déjà conclu un protocole à l'Automne 2017 en vue de formaliser les échanges d'informations sur les agents qui relèverait successivement de l'une ou de l'autre, et donc pour ces 2 raisons, c'est de réserves l'avis défavorable et en cohérence la vie sur les sous-amendements est aussi défavorable. Nous allons passer au vote, donc on commence par le sous-amendement numéro 28 à monsieur Bigot non je sur l'amendement lui-même, donc, qui, pour l'amendement numéro 28.

nous, nous ne sommes pas favorables à cette à cet amendement parce que on commence à faire une confusion sur les missions de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la Haute autorité saisie je rappelle à la tête, c'est actuellement été créée pour contrôler la situation des membres du gouvernement, des élus, nous-mêmes, ici présent, etc, des élus locaux, si l'on souhaite effectivement qu'elle puisse aller au-delà et le fait déjà pour la haute fonction publique avec des un certain nombre de déclarations pour Léo magistrats etc, il n'y a aucune raison que les contrôles relatifs à ces personnes soient soumis à d'autres cas, ceux de la Haute autorité, elle-même, donc je ne comprends pas très bien pourquoi on veut complexifier les choses en en rajoutant au sein de la Haute autorité, une commission spécialisée qui est composé de manière différente, il n'y a aucune raison de le faire et c'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas cet article additionnel après l'article ce que 5 malgré l'avis favorable de la commission. Donc nous passons au vote de cet amendement 16 rectifier qui est pour.

D'accord, bah Tobler vous avez la parole merci. Cet amendement vise à une une clarification du positionnement institutionnel de la commission déontologique qui est pour l'heure, placé auprès du 1er ministre l'exigence d'indépendance inhérente à ces travaux et le fait que la Haute autorité pour la transparence de la République soit devenue une agence ministre ne tiennent sera-t-il indépendante en 2013 plaide pour ce genre changement de statut, cet amendement et Éric donc la commission de déontologie de la fonction publique à l'autorité administrative indépendante, cette transformation est un 1er pas vers une fusion entre la haute autorité administrative haute autorité pas transparent les publics autre mesure proposée dans ses rapports, dans un souci de clarification et de simplification du cadre déontologique dans la sphère publique. L'avis de la commission Madame Coste

Merci monsieur le président, le gouvernement constate que votre moment est satisfait ne signifie pas qu'il approuve sa satisfaction, mais le constat, donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. nous allons passer au vote qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est rejeté, nous passons à l'article 6 le 11 rectifier. Monsieur Artano vous avez la parole. Merci monsieur le président, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement très important et là encore, qui ne relève pas du gadget on lisant l'étude que sont les énarques devenus, nous avons été stupéfaits découvrir que certains d'entre eux passent plus de la moitié de leur carrière dans le secteur privé, tout en conservant leur statut d'agent public, nous avions en 1er lieu visé les détachements, alerté par le laconisme de la loi qui dispose, je cite, que les détachements peuvent être de courte ou longue durée, les travaux de Josiane Costes ont montré que le régime juridique utilisée pour le pantouflage est actuellement principalement la disponibilité, ce qui nous a permis de réajuster ses dispositions, il nous semble que cette situation mérite une clarification et le sait, s'il passe par la définition de délais légaux pour les disponibilités de pantouflage que nous proposons de fixer à 5 ans sur la base de la promesse de campagne du président Macron quelle est la frontière entre le secteur public et les secteurs privés si des agents publics peuvent construire des carrières dans le secteur privé, sans jamais avoir rejoint de l'administration, le maintien anormalement long de fonctionnaire en disponibilité entraîne une réelle difficulté, en matière de gestion des ressources du Maine puisque théoriquement, ces agents publics ont vocation à réintégrer leurs services, en outre, on peut facilement juger que la réussite de leur intégration sera inversement proportionnel à la durée passée dans le secteur privé, c'est pourquoi nous vous proposons cet amendement qui veille spécifiquement à ne pas viser l'ensemble des disponibilités en raison de celles décidées d'Office sur le fondement de raisons familiales ou encore de recherche, nous avons également pris garde dans notre rédaction à ce qu'elle n'allonge pas la durée des délais actuellement prévus, ou encore de création ou de reprise d'une entreprise 2 ans actuellement. La commission a beaucoup discuté sur cet article, la mise en disponibilité d'un fonctionnaire est toujours limitée dans le temps, quel qu'en soit le motif, par exemple la mise en disponibilité pour création d'entreprise est limitée à 2 ans non renouvelable, elle n'est accordée que sous réserve que l'activité envisagée soit compatible avec les activités exercées dans le secteur public au cours des 3 années précédentes, les autres cas mise en Libye, en disponibilité ne répondent pas aux mêmes critères de durée ni de compatibilité par conséquent le principe posé par le président le présent amendement, nul ne peut se maintenir indéfiniment en disponibilité et déjà satisfait en outre la durée proposée pour une mise en disponibilité pour exercer une activité lucrative serait plus favorable que le droit en vigueur, ce qui semble contraire à la volonté des auteurs, donc c'est une demande de retrait de la commission des lois, ou à défaut un avis défavorable de la commission des lois. Merci la vie du gouvernement. Merci Monsieur le Président, c'est, c'est le même avis pour exactement les mêmes raisons.

Je vous sur Monsieur le Monsieur le Président, vu le sort qui a été réservé à mes amendements sont toutes bien anodin. J'ai quand même conscience que je n'ai absolument aucune chance, donc je ne ferai pas perdu notre temps. Donc le suivant aussi très bien l'avis de la Commission sur c'est peut-être vous allez être plus long que lui. Pour les 2 amendements les amendements même de 3 procède de la même philosophie, limiter le nombre de fonctionnaires appartenant à un même corps qui serait en même temps en disponibilité de la fonction publique, donc s'étonne : demande de retrait ou à défaut un avis défavorable pour les 2 amendements. Très bien, donc, le gouvernement dit quoi.

C'est pour quand même l'élément pour qui est contre qui s'abstient, c'est le même vote pour les 2 amendements. Donc nous passons après l'article 6 le 9 rectifier bis. Monsieur Artem dont vous avez la parole. Merci monsieur le président, merci à mon collègue Colomba de nous donner un peu de temps cette PPL en l'état du droit, rien ne prouve que les avis de compatibilité ou de compatibilité avec réserve la commission déontologie sont respectés par les fonctionnaires pendant leur pantouflage dans le secteur privé, le récent rapport de nos collègues députés Fabien Matras, c'est Olivier Marlex souligne d'ailleurs comme matière de contrôle des avis des éventuelles réserves, il convient de rappeler que la commission de déontologie ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle a posteriori pas même d'un droit d'interroger les agents partis dans le privé, sa proposition numéro 9 vise en ce sens à contrôler dans la durée, le respect des réserves au travers d'une interrogation annuel des personnes interrogées et leurs employeurs, par la commission de déontologie le présent amendement reprend cette proposition tout on la circonscrit vont aux postes de fonctionnaires les plus sensibles, il reprend, pour ce faire, le périmètre des déclaration de situation patrimoniale des fonctionnaires ont employes dans le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions ne justifie mentionnées sur une liste établie par décret en conseil. Merci l'avis de la commission Madame Coste. Merci Monsieur le Président, c'est un avis favorable. L'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, il faut d'abord rappeler que, conformément à l'article 35 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées au fonctionnement de la commission déontologique, la vie de ladite commission, et la décision de l'administration sont transmis à l'entreprise ou à l'organisme qui a accueilli l'agent concerné, l'entreprise est donc déjà en mesure de savoir si le fonctionnaire qui a rejoint ou non respecter l'avis de la commission, par ailleurs, cet amendement déposé le suivi du respect des obligations déontologiques émise par la commission par les entreprises qui ne nous paraît pas souhaitables cette charge administrative supplémentaire serait d'ailleurs de nature à les dissuader de recruter des agents publics et par voie de conséquence, interrompent sac à la mode à la mobilité des carrières entre public et privé, telle que souhaitée par le gouvernement, c'est à l'administration d'origine, en lui-même, de s'assurer du respect des obligations déontologiques sous peine pour les gens concernés de sanctions disciplinaires, au pénal, donc, pour ces raisons, l'avis défavorable. Il y a, il y a un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté, nous passons à l'article 7 avec un amendement numéro 27 de la commission Madame Cosse. C'est simplement un amendement de coordination. Eh bien le gouvernement bon qui est pour. Qui est contre, il était adopté, on passe au vote de l'article 7 qui est pour. Qui est contre elle est adoptée après l'article 7 Monsieur Collombat 25 rectifier bis. C'est un autre problème c'est, comment dire, la capacité d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, donc de remplir plusieurs fonctions, à la fois. on s'en était étonné d'ailleurs, je me rappelle quand on avait fait la mission, la mission d'enquête sur les hautes autorités sous la présidence de Jacques Mézard, on s'était étonné de la capacité de certains être partout.

je vous lis simplement je me réfugie derrière une autorité puisqu'il s'agit quand même de Jean-Louis Debré, c'est pas rien, il est parlant. Une référence, comment se fait-il qu'en magistrats, dont la fonction est d'être conseil du gouvernement puissent être rémunérés en plus comme conseil d'une administration ou d'un établissement public qui, en outre, dispose déjà d'une direction juridique ce cumul est insensé, non. Eh ben apparemment non. Madame votre avis au dos de la commune. Merci Monsieur le Président, cet amendement propose de s'inspirer des incompatibilités parlementaires pour interdire, fonctionnaire ou agent public d'exercer activité de conseil le cumul d'activité déjà soumis au contrôle de la commission d'déontologie de la fonction publique, en application du grand 2 de l'article 25 oct et c'est du grand 3 de l'article 25 cepté de la loi du 13 juillet 1983 il n'est donc pas indispensable de prévoir une interpellation générale et absolue, c'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis, un avis défavorable de la commission des lois. Monsieur le Ministre votre avis. Comme l'a dit Madame le rapporteur, l'ensemble des agents publics sont concernés par l'application des dispositions de la loi de 1983 ainsi que les dispositions du décret du 27 janvier 2017 interdire spécifiquement le cumul d'activité pour les grands corps nous sommes crée une situation juridiquement fragile, au regard du principe d'égalité donc l'avis défavorable.

Merci Monsieur le Président, cet amendement, déjà adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie publique, numéro 2000 17339 du 15 septembre 2017 vise à prévenir l'utilisation afin lucrative d'un réseau d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d'une mission de service public en introduisant un délai de 3 ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public pour rendre à César ce qui est à César, il faut préciser que cet amendement avait été déposé par le sénateur gêné lors de l'examen de la loi sur la confiance, nous avons pris la liberté de le déposer en considérant qu'il s'insérer bien dans l'esprit de notre proposition de loi et afin de renforcer sa nature consensuelle. La commission le la vie de Madame Coste. Merci monsieur le président, un ancien fonctionnaire qui souhaiterait créer un cabinet de conseil après avoir démissionné de la fonction publique doit saisir la commission déontologie de la fonction publique qui doit s'statuer s'statuer sur la compatibilité des nouvelles fonctions qui serait exercée dans le secteur privé avec celles qui le seront dans le secteur public aussi, après y avoir de nouveau réfléchit y avoir débattu la Commission appelle finalement jugé préférable de son tenir auprès des actuels pour le moment, plutôt que de substituer au contrôle actuellement exercées par la commission de l'anthologie une interdiction totale, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, tempère renforcer davantage ce contrôle pouvoir de prévoir une interdiction générale, laissant à ce dispositif de contrôle, le temps de produire leurs effets, donc la commission Allemagne un avis défavorable. Très bien monsieur le ministre, votre avis. Merci Monsieur le Président, l'avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le maire appartenant. Merci. Qui est pour.

Aucun la même ligne que le précédent, et que le suivant cette amène cet amendement également adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie politique vise à interdire aux anciens fonctionnaires ou agents publics indisponibilité et il y a exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée aux pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d'activité pendant un délai de 3 ans, il avait également déposé par monsieur Très bien, donc on, on dit que c'est les 2 amendements suivants 14. Non, on va, on va les faire séparément Madame Coste. Merci monsieur le président, donc c'est la même philosophie que l'homme que l'amendement précédente donc la commission des lois a émis un avis défavorable.

qui est contre.

Cet amendement également adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 vise à limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d'intérêts au préau ou pour le compte d'une personne morale de droit public et dont ils auraient fait partie, comme les 2 précédents, c'est le produit monsieur jeunesse. Très bien, madame la rapporteure. Une file monsieur le Président, même philosophique pour les précédents donc la commission a émis un avis défavorable. Monsieur le Ministre.

Non, il est rejeté d'une voix il y a mais bon des votants changé entre-temps temps et tout, mais c'est comme ça, on va passer à l'article 7 après l'article VII, le 26 rectifier. Et c'est le dernier amendement Monsieur Collombat. En demandant reprend une disposition que le Sénat à l'unanimité a voté par 2 fois. Il est ici parce que le sort réservé. Aux élus locaux. Touché quand ils sont touchés par

Donc je pense que vu les précautions comprend pas perturber les gens qui risque d'être en situation de conflit d'intérêts pourrait profiter aussi un peu aux élus locaux qui se voit reprocher des prises illégales d'intérêts parfaitement fictives, donc il s'agirait simplement de remplacer la définition actuelle, c'est-à-dire un intérêt quelconque par un intérêt personnel distinct de l'intérêt général, donc évidemment exclu tout problème personnel etc, mais au moins ça serait plus clair, voilà, ça fait 2 fois que le Sénat, le vote. Il n'y a été donné aucune suite à l'Assemblée nationale, je m'étonne de ce cette dualité de de traitement. Eh bien, madame la rapporteure va donner son avis. C'est un avis favorable. Ben voilà monsieur Colomba vous êtes pas venue pour rien monsieur le ministre, à votre avis. Merci Monsieur le Président, l'avis est défavorable, défavorable car nous considérons que la proposition de loi et malgré les réserves

Le la parole à à monsieur le président, pour sur cet amendement. Monsieur le ministre, je suis très déçu de votre prise de position et nous avons l'expérience. Dans nos départements, avec les maires, au contact duquel nous sommes quotidiennement de trop nombreuses difficultés d'application de la législation pénale en matière de confiner la notion d'intérêt quelconque. A été étendue à la prise en considération d'intérêts qui peuvent être caractérisées par de simples relations amicales ou familiales Direct voir l'appartenance à des eaux socia Sion à but non lucratif qui rendrait pénalement sanctionnable un élu qui aurait participé à une décision publique et qui aurait tout simplement des Liens tout à fait conforme d'ailleurs à ce qu'on peut te attendre d'un engagement au service de la vie sociale et de la vie de la collectivité avec des structures qui ne représente aucun intérêt d'argent il faut que cela cesse et notre collègue Pierre-Yves Collombat avec beaucoup de persévérance, le débat mais nous le faisons aussi nous-mêmes dans d'autres circonstances, à chaque fois que nous pouvons le faire, j'entends bien que ça n'est pas le bon support mais reconnaissez tout de même Monsieur le Ministre, que cette question devient lancinante, vous devez savoir que beaucoup d'élus locaux sont découragés que beaucoup d'élus locaux se sentent contraints dans leur action, service de l'intérêt général, par une accumulation de réglementations et de risques judiciaires qui sont tout autant d'entraves au service de la population hé bien puisque nous avons l'occasion de le faire, votons cette disposition mais ne la votent aurions avec une satisfaction d'autant plus grande que le gouvernement montrerait un peu d'attention aux élus de notre pays en acceptant cet amendement. Bon le le ministre a demandé la parole, mais peut-être très fertile parler après tout ceux qui ont demandé la parole, donc Monsieur Hervé. Monsieur, Président de sionisme chaque collègue je vais pas m'étendre mais je rejoins complètement la position du président de la commission des lois a merci Pierre-Yves Collombat d'avoir déposé cet amendement je crois finalement pour la 3ème fois je ne doute pas qu'il soit adopté, pour vous dire Monsieur le ménisque on peut distinguer 2 choses : d'abord la réflexion globale sur le statut des élus locaux, qui est une réflexion qui a été engagé ces jours-ci par le Sénat, notamment par sa délégation aux collectivités territoriales qui est suivie de près au sein de notre commission des lois et qui est une question de fond, mais la question de l'amendement Colomba que nous examinons cet après-midi,

qui n'est pas dans mon département et où le le maire d'une commune rurale, avocat de son état, a assuré la défense de sa collectivité et a été condamné pour prise illégale d'intérêt, au profit de la réputation qu'il aurait pu potentiellement tiré de l'affaire qui l'a lui même défendu en faisant en faisant cela, il a défendu sa collectivité, c'est quand même le rôle d'un maire, il a été il a été habilités par le conseil pour le faire, il ne il n'en a tiré évidemment aucune rémunération, il a fait faire des économies et cette petite commune rurale et il a été lui-même condamné pour prise illégale d'intérêts audits de la femme a comme on dit en latin la réputation qu'on aurait pu tirer de cette affaire, ça devient quand même fâcheux ça alimente le discours à l'égard des élus locaux qui tirait de d'un profit quelconque de leur mandat et je sais que monsieur, mais vous êtes très attentif à cette question : ne tardez pas trop à intervenir sur ce sujet, je crois que on ferait les uns les autres oeuvre utile. Cet amendement qui a toute sa pertinence, même s'il n'a peut-être pas sa place dans cette loi, mais il faut bien qu'il des articles dans cette loi est très révélateur très révélateur de la manière dont, à un moment donné, on a été capable, dans les années 92 93 je me souviens qu'il était au gouvernement de faire des textes de loi au nom de la transparence pour éviter la corruption etc qui qui aboutissent aujourd'hui dans la jurisprudence parce que c'est des instruments que l'on donne à la justice qu'il applique des interprétations qui se retourne contre les élus et qui ne vont pas dans le sens qu'on veut, cela à l'heure où on a qu'on est en train d'aborder un texte de nouveau sur les confiner intérêt devrait nous amener à beaucoup de modestie, sur la manière dont on doit légiférer en la matière et où parfois on a des textes qui se retourne et qui n'ont pas le but que l'on avait l'amendement de Pierry Colomba doit être votée en l'état, parce que c'est un amendement d'appel ça l'amendement d'appel, monsieur le ministre, quand vous nous dites que ça n'a pas sa place ici, dites à Madame la Garde des Sceaux, que ça vaut le coup de maître dans la place, des textes de droit pénal qu'elle veut nous soumettre dans peu de temps, ça serait intéressant que le gouvernement de ce point de vue-là sont attentifs à la situation dans laquelle se retrouver quelques élus locaux. Monsieur Colomba : c'était le dernier amendement

trouvez-vous normal que quelqu'un qui représente qui représente sa sa commune dans une association locale parce que la commune est membre de droit du comité machin ou je sais pas quoi puisse être inquiété, si d'aventure il a oublié de sortir

Non mais on c'est complètement loufoque, si vous ne le savez pas ben on vous l'a dit bon donc voilà c'est alors en plus quand on voit le traitement de faveur Sajid 100 alors là du haut fonctionnaire

Monsieur Mohamed, dit monsieur le président, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, j'ai tout à l'heure, expliquer quelle était la position de mon groupe, par rapport à cette peine, mais je voulais vis-à-vis de cet amendement et à titre personnel, en cohérence avec moi-même, en cohérence avec mon vote intérieure à la commission des lois, personnellement, je voterai c'est amendement. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci monsieur le président, rassurez-vous, ce sera bref il sent Monsieur le Ministre, que nous serons invités prochainement examiner un projet de loi dit pour une société de confiance, hé bien cette confiance, Monsieur le Ministre, je vous invite à l'exprimer avec tout votre gouvernement en 1er pour les élus locaux pour les mères, parce que ce sont eux qui tiennent encore ce territoire ce pays à peu près ensemble vous avez cette belle occasion de nous aider à pousser cet amendement auprès du gouvernement, peut-être sous une autre forme dans un meilleur véhicule mais en tout cas fait confiance aux élus locaux, vous ne le regretterez pas Monsieur le Ministre. Eh bien, devant tous ces appels pressants, mais non, monsieur le titre va parler et va vous répondre. Quelques mots Sydney président pour pour répondre et d'abord dire au président que j'merci madame de La Gontrie je j'apprécie toujours votre sollicitude et je pense que j'aurais pu vous renvoyer à peu près le même compliment sur les explications qu'a données le président bah, j'aurais pu reprendre à mon compte, chacun des mots, vous avez prononcé Monsieur le Président et j'aurais pu les reprendre à mon compte parce que, en écho à ce que disait monsieur pas un instant des élus locaux, j'en connais, j'en suis en en j'suffisant et j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance de président association qui rassemble les élus 2002 2500 à 25000 habitants, avec beaucoup de ses adhérents, confrontés à cette difficulté je vais plus loin dans cette explication pour vous inviter à regarder ou en tout cas à retrouvez le compte rendu de la commission des lois de l'Assemblée nationale du 18 juillet dernier au cours de laquelle nous avons examiné le projet de loi pour la confiance dans la vie politique et j'avais dit à Madame la Garde des Sceaux, les difficultés qui sont posées par la définition actuelle de la notion de crise illégale d'intérêt avec les mêmes arguments que ce que vous avez évoquées, je maintiens, je persiste à dire que cet amendement n'a pas sa place dans un texte sur la déontologie en matière de fonction publique, et pour ce qui concerne Léo Léo fonctionnaires tout particulièrement donc l'avis du gouvernement reste un avis défavorable, mais je puis vous assurer que je serai relayer les préoccupations qui sont les vôtres, auprès de Madame la Garde des Sceaux, que si je ne fais pas moi-même et me semble que ce sera fait encore plus directement parce que nous partageons cet objectif-là et je souhaite que les prochains textes qui seront soumis à votre approbation ou en tout cas à votre examen par la garde des Sceaux, puisse nous permettre collectivement de déboucher sur ce problème-là, en l'état par cohérence, c'est parce que nous considérons que ça n'a pas sa place dans ce texte, la vie reste défavorable mais vous notez que le gouvernement sera attentif à tout cela.

Qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité, c'est une bonne façon de finir l'examen de ce texte, je demande s'il y a des explications de vote sur l'ensemble du texte Monsieur Bigot. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense que pour le groupe RDSE, qui est à l'initiative de cet texte doit avoir une grande, une alors qu'il y avait une forte volonté d'amplifier la déontologie en fonction publique, on arrive à un texte qui a quelques articles qui sont maintenus. On a un rapport parlementaire, porté notamment par un membre de en marche, qu'il fera des propositions d'ailleurs accompagné d'une étude d'impact, comme l'indique le Conseil d'État en disant vérifiant aujourd'hui ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas c'est la confiance de nos concitoyens. Notamment dans la haute fonction publique et cette confiance est entamée. à mon sens autant. à l'égard des élus et des parlementaires rançon et que il faudra bien effectivement à un moment donné, que l'on sache comment on peut rétablir cette confiance sans imposer, d'ailleurs, la haute fonction publique et les élus, y compris ceux qui siègent au gouvernement, comme ça a été dit dans cet article du Monde, donc je pense aujourd'hui que ce texte contient d'articles qui sont pas inintéressants, c'est une proposition de loi qui n'ira sans doute pas loin, c'est une proposition de loi qui contient quelques appels utiles : celui qui vient de trophées et dans d'autres domaines. Donc je pense que notre groupe va simplement s'abstenir pas voter contre mais parce qu'il y a une trop forte attente par rapport à ce qu'il faut faire mais qui nécessite plus qu'une simple proposition qui nécessite, monsieur le ministre de la part du gouvernement, une vraie étude d'impact de vraies propositions qui peuvent s'inspirer notamment du rapport qui a été fait par les députés, j'ai d'ailleurs constaté que sur l'une des propositions de ce rapport, la proposition numéro 9 vous aurez constaté que le gouvernement n'a pas d'amener d'avis favorable, j'espère au moins que pour une fois en marche se rate entendu. Merci monsieur Laménie, vous avez demandé la parole pour l'explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, famille, chers collègues, au très rapidement parce que je crois qu'il y a eu une participation active, elle mérite revient naturellement aux auteurs au niveau du groupe RDSE et et je crois qu'on on a pu faire des avancées faire avancer aussi des sujets qui ne sont pas simples pour les serviteurs de l'État, servir l'intérêt général, c'est vrai, au quotidien, puis de l'autre côté, ben les amendements qui ont été examinés et puis je crois que le travail collectif, au fait par les collègues le mérite revient aussi aux collègues de la commission des lois, et on a pu mesurer, notamment sur le dernier amendement ont la qui fait un parallèle avec l'engagement des élus locaux, tout confondu, quelle que soit la taille des communes, c'est aussi un engagement de servir du service public au service de nos concitoyens, quelle que soit la taille des des des villes, villages et bourgs et je crois que c'est aussi un engagement et puis le parallèle avec la mission d'élus, d'engagement pour les autres,

Donc encore plusieurs interventions Monsieur Collombat. de l'objet de de nos débats de d'aujourd'hui, je peux vous. Simplement vous dire que j'aime, on nous ne pouvons pas laisser penser qu'on a fait même un pas vers l'amélioration de cette situation, cette situation est grave qu'on ne voulait pas voir, on veut pas voir et je constate que les défenseurs et les pantouflards et les amateurs de Porto tournantes sont enfin ah ça va pas se passer comme ça et je ne pense pas que ça se sache, ça se passe par des petits bouts d'amélioration de la de la législation de la déontologie, etc, il y a un problème de fond, un problème structurel qu'-ce que que devient notre République,

Merci le Monsieur présent pour l'équipe, situation de voter et donc la position du groupe de Lyon centriste d'abord pour remercier nos collègues du groupe RDSE pour cette préfiguration du grand débat qui va nous emmener dans quelques mois, à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur cette question de de la fonction de la fonction publique en général, pour vous dire, Monsieur le Ministre, que déjà le le Sénat dans son rôle pour les parlementaires anticipées ce ce grand chantier qui est la qualité des débats cet après-midi à démontrer que, il y a des sujets rejoins en partie ce vient à notre collègue Pierre-Yves Collombat pour dire que, effectivement, dans la confiance entre nos concitoyens et leurs dirigeants et leurs dirigeants publics et parmi les dirigeants publics et aux fonctionnaires, il y a nécessité à ce que des modifications soient faites sur un plan symbolique, on l'a déjà fait avec les élus, on pourrait le faire et aux fonctionnaires, mais aussi sur le plan du statut, sur l'organisation même de la fonction publique dans notre pays qui a nécessité à évoluer, c'est pour que la raison pour laquelle le groupe Union centriste a participé à ces débats soutenu un certain nombre d'évolution du texte et votera favorablement à cette Merci monsieur Léonard. je ne sais plus si c'était Trotski ou si c'était Lénine qui disait qui disait un pas, un pas en avant, un pas en avant Lénine merci, un pas en avant vaut mieux que mille programmes voilà simplement ce que je voulais vous dire.

Vous voulez moi non 10 minutes.

La séance est reprise, il reste dans cette niche parlementaire jusqu'à 18 heures 37 donc il y a le temps. La science et donc reprise lors du jour appelle la discussion de la proposition de loi sur le régime de l'exécution des peines, des auteurs de violences conjugales, présenté par Madame Françoise Laborde et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe RDSE. Dans la discussion générale, la parole et donc à Madame Françoise Laborde, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que j'ai souhaité déposé avec le soutien de la grande majorité des membres du groupe RDSE a pour objet d'aborder les problèmes rencontrés dans l'application et l'aménagement des peines prononcées à l'encontre des auteurs de violences conjugales et de tenter d'y apporter une solution, les circonstances qui m'ont conduite à prendre cette initiative, sont à la fois le résultat d'une réflexion personnelle engagée sur le fond dans le cadre des travaux de la délégation droits des femmes, dont je suis membre, depuis mon élection au Sénat en 2008, mais aussi le fruit de rencontres avec les acteurs associatifs dans mon département, la Haute-Garonne, j'ai été alertée par un collectif associatif sur l'incompréhension des victimes de violences conjugales et de leurs familles face aux conséquences de certaines décisions judiciaires en matière d'aménagement des peines les 2 faits relatés pose le problème dans son ensemble et nous interroge un homme peut-il être placé derrière les barreaux pour de menus trafics de stupéfiants, alors qu'un autre et placé en liberté surveillée, quand il est attesté par une décision judiciaire qu'il a à plusieurs reprises frappé violemment sa compagne, si l'on peut comprendre la démarche des juges d'application des peines qui autorise ces aménagements, on ne peut rester sourd à la détresse des familles et sous un mouvement des enfants qui voient le bourreau de leur mère, laissée libre suite à une décision de justice qui l'a pourtant reconnu coupable le poids symbolique de cette pratique est extrêmement lourd de conséquences, c'est un contre-signal adressé en matière de Lille, lutte contre les violences conjugales, on objectera peut-être que ma proposition risque d'aggraver le phénomène de port de surpopulation carcérale les lieux privatifs de liberté sont surchargés et la restriction des aménagements de peine aurait directement pour conséquence une augmentation de ses effectifs, mais il s'avère que les violences conjugales sont très spécifiques, elle se caractérise par un dénominateur commun à l'auteur des faits, comme à la victime, je veux parler du déni, nourrie par le phénomène de l'emprise c'est une carrure caractéristique constante dans ce type de délit. Le législateur ne doit perdre de vue ni cette particularité, ni la question de l'avenir des enfants qui sont souvent pris au piège dans des situations délétère pour leur construction et qu'il nous faut protéger trop souvent, ils sont les premiers témoins otages et malheureusement victime collatérale prise dans les mailles des violences conjugales, la réponse judiciaire est-elle appropriée face à ces violences particulières, c'est la question que j'ai voulu soulever aujourd'hui dès qu'il y a violence les institutions doivent réagir à la mesure du problème car laisser ces violences installé dans l'intimité des couples, c'est laisser le phénomène s'aggrave en fréquence et en intensité, certains experts ont même proposé de supprimer les mains courantes en cas de violence conjugale, car elle donne le signal aux victimes que leurs plaintes, mais ni prise au sérieux ni suivi d'effet je ne suis pas allé jusqu'à cette extrémité dans ma proposition de loi mais j'ai entendu les conseils de juges expérimentés, l'arsenal juridique dont nous disposons, sous-estime la prise en charge des auteurs de violence qui devrait se faire en amont d'Airbus dès les premiers signalements, j'ai choisi de déposer cette proposition de loi pour pointer l'inadéquation des mesures alternatives à la privation de liberté au cas de violence conjugale, à fortiori au cas d'emprise et nous conduire à nous interroger collectivement sur des situations concrètes insupportables auxquelles sont confrontées les victimes et leurs familles, comment s'assurer que ces aménagements de peine ne soit pas prononcé lorsque la liberté surveillée expose les victimes ou leurs familles à de nouvelles violences nos magistrats sont-ils suffisamment formés pour déceler les phénomènes d'emprise pour tous sans certaines victimes a demandé elle-même la remise en liberté de leurs agresseurs, autant de questions sans réponse, si je comprends la démarche des juges d'application des peines qui pour prenons ces aménagements dont je n'ignore pas les raisons, je considère que le législateur ne peut rester sourd à la détresse des familles des victimes, c'est la raison pour laquelle mon texte prévoit d'exclure des dispositifs d'aménagement des peines, notamment à Binic sur les auteurs de violences conjugales, afin de les maintenir à distance de leurs victimes, pour autant, j'ai bien entendu les réserves juridiques exprimées par nos collègues de la commission des lois et je suis sensible à leurs arguments, l'article 1er aurait pour conséquence d'empêcher le prononcé de certaines mesures probatoires encadrant les sorties de détention alors que celle-ci pourrait réduire le risque de récidive quant à l'article 2 les membres de la commission des lois ont estimé qu'il porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, je peux l'entendre mais c'est aussi à la loi, de mettre en place les moyens de sortir du cercle infernal des violences pour protéger les victimes et actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas, je cite le rapport de la commission sûrement texte le Champ d'application de ces dispositions apparaît d'illégal gravité contrairement à celui des infractions terroristes dont les auteurs font l'objet d'un régime dérogatoire d'exécution des peines, tout est question en effet d'appréciation de la gravité du Champ d'application et même si je ne mets pas sur le même plan Terrorisme et violence conjugale, l'ampleur de ce fléau dans notre pays me semble suffisamment vaste pour être considéré comme relevant d'une forte gravité notre responsabilité face aux victimes et collective, je vous en rappelle le contexte global en quelques chiffres, ces 10 dernières années, le bilan des violences au sein des couples en France est toujours aussi implacable dans un rapport récent, la délégation droits des femmes du Sénat rappeler qu'entre 2006 et 2016, ce sont 1200 femmes qui sont mortes sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire intime soit un meurtre sur 4 commis en France, les violences au sein du couple reste donc un fléau une réalité cruelle, en dépit de la mobilisation des services publics et du renforcement du cadre législatif, plus de 223000 femmes sont encore victimes de violences conjugales, chaque année, ce chantier devrait être engagée dans le cadre de la loi Justice à venir que vous viendrez nous présenter dans les prochains mois, Madame la Ministre, parmi les 5 axes de réforme annoncées, celui du sens et de l'efficacité des peines à retenu toute mon attention, c'est bien de ce dernier chantier dont relève mal proposition, elle y a toute sa place, elle pourrait peut-être également trouvé un écho favorable dans le nouveau projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles qui sera prochainement soumis au Parlement à la veille d'une réforme judiciaire et d'une loi contre les violences sexistes et sexuelles, je comprends bien que le texte de ma proposition de loi ne satisfait pas les juristes les plus émérites de notre assemblée, mais j'espère néanmoins que mes arguments vous auront convaincu de faire évoluer ces questions mais chers collègues dans les véhicules législatifs qui conviendra et conformément à la proposition et à l'esprit de ma proposition de loi, c'est-à-dire renforcer l'efficacité des peines alternatives de façon la plus adaptée possible aux spécificités des actes de violence envers les femmes dans les situations d'emprise conjugale d'expérience, je sais qu'il peut être nécessaire de déposer une proposition de loi pour soulever un débat de société et faire bouger les lignes, je vous remercie. La parole est à madame Brigitte Lherbier, rapporteur de la commission des lois à la 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, ce président, chers collègues, la proposition de loi présentée par Madame Françoise Laborde propose la création d'un régime dérogatoire en matière d'exécution des peines applicables aux seuls auteurs de violences conjugales, c'est un peu ce qui ne gère ces derniers seraient exclus de l'attribution de crédits de réduction de peine les personnes incarcérées pour ces violences ne pourrait également plus sollicité une suspension ou une ou un fractionnement de leur peine pour un motif grave d'ordre médical, familiale, professionnelle ou sociale, enfin, ces personnes ne pourraient plus bénéficier de mesures de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. Cette proposition de loi vise ainsi appliquer le régime dérogatoire, créé par la loi du 3 juin 1000 2016 applicable aux personnes condamnées terroriste aux auteurs de violences conjugales. Nous partageons tous, ici, chers collègues, l'objectif d'améliorer la lutte contre les violences conjugales, bien sûr, adjointe à la sécurité, Tourcoing, vous savez, j'ai été confronté aussi à ces horreurs régulièrement Madame mais il faut avant tout être efficace. Pour cette raison, la commission des lois n'a pas adopté cette proposition de loi en raison de nombreuses difficultés juridiques, vous l'avez évoqué et pratique qu'elle présente. Nous ne voulons pas céder à la démagogie, vous non plus, je suppose, nous essayons d'être rigoureuse, c'est l'essence même du Sénat du travail au Sénat n'est-il pas en 1er lieu le Champ des infractions retenues pour l'application du régime dérogatoire poser question. Tout d'abord, il recouvre des violences d'inégale gravité par exemple l'homicide par conjoint n'est pas visé, alors qui est inclus le délit d'appels malveillants. Deuxièmement, il concerne des infractions qui ne peuvent par définition être commises à l'encontre d'une victime par son conjoint par exemple sont visées certaines infractions pénales uniquement constituée lorsque les violences exercées en groupe, je pense au délit d'embuscade ou encore de bandes organisées. La commission des lois n'a pas adopté cette proposition de loi car il serait incohérent et contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, d'exclure les seuls auteurs de violences conjugales du bénéfice des crédits de réduction de peine. Et aussi de la possibilité de voir leur peine aménagée dans un centre de semi-liberté par exemple l'comme évoqué cette proposition de loi s'inspire du régime dérogatoire applicable en matière de terrorisme. Néanmoins, ces dispositions applicables en matière de lutte contre le terroriste semble difficilement pouvoir être être étendue aux chants des infractions retenues par la proposition de loi qui recouvre des comportements, je disais tout à l'heure d'inégale gravité certaines infractions visées ne sont. sont. Que on ou d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende à l'inverse, les infractions terroristes sont au minimum puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et au maximum de la réclusion criminelle à perpétuité, cela n'apparaît pas comparables. Surtout, le, le, la commission de lois, d'autre part estimé que cette proposition de loi serait contre- productive pour l'objectif recherché par exemple l'article 1er propose de réduire les mesures d'aménagement pouvant être proposés aux condamnés déjà incarcéré. Or, a fortiori dans un cas de violence conjugale, il est nécessaire d'éviter les sorties sèches et d'accompagner les libérations de condamnés incarcérés par des mesures probatoires. Les suivi probatoire permettent d'obliger les condamnés à suivre des traitements à se soigner à ne pas rencontrer la victime à être entendu par des groupes de parole, nous avons eu l'occasion d'échanger avec eux des magistrats en audition. Enfin, la proposition de loi ne semble pas correspondre au problème soulevé aucune disposition n'est proposée pour modifier la possibilité pour le tribunal correctionnel d'aménager à Benicio au stade du jugement, les peines d'emprisonnement prononcée dès le stade du jugement, le tribunal correctionnel peut en effet aménager une peine d'emprisonnement on a placement sous surveillance électronique ou une mesure de semi-liberté, aucune disposition n'est proposée pour modifier la procédure d'examen systématique par le juge d'application des peines en vue d'un aménagement des peines d'emprisonnement, d'une durée inférieure ou égale à 2 ans des condamnés dès Nona car c'est cette procédure qui est en réalité très, très, très critiqué cette proposition de loi ne changeraient donc en rien au constat de non-exécution des petites peines d'emprisonnement que ça soit dans ce cas là où d'autres, aucune disposition n'est proposée pour modifier la possibilité pour le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines de prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique, en application de l'article 723 tiré 7 du code de procédure pénale, or je rappelle que le Sénat a déjà adopté plusieurs réformes d'envergure du régime d'exécution des peines, madame la Ministre, peut peut-être s'en inspirer et nous reprendrons ce travail quand vous le souhaitez, avec vous, Madame la Ministre, en janvier 2017, le Sénat a adopté la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale présenté par messieurs François-Noël Buffet et Bruno Retailleau. Son article 20 à supprimer le principe de l'attribution automatique des crédits de réduction de peine pour tous les condamnés détenus et en conséquent bleu régime actuellement prévu pour des réductions supplémentaires de peine tués un du Code de procédure pénale, qui deviendrait le seul régime de réduction de peine, c'est notre façon de de voir les choses surtout en n'octobre dernier, le Sénat a adopté la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présenté par notre président de la commission des lois, Philippe Bas, son article 27 prévoit la suppression de l'obligation d'examen par le juge de l'application des peines avant mise à exécution de toutes les peines d'une durée inférieure ou égale à 2 ans d'emprisonnement ou un an, en état de récidive légale, cette mesure permettrait de répondre à la légitime incompréhension des victimes dont vous parliez tout à l'heure Madame ou des proches des victimes, de ne pas voir incarcérer une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de 18 mois vous l'avez évoqué tout à l'heure. Beaucoup de choses doivent encore être faites pour améliorer la protection des victimes de violences conjugales, je suis tout à fait d'accord avec vous Madame Laborde, notamment en généralisant le dispositif Tél grand danger par exemple. Ou en main, encadrant le dépôt de plainte, néanmoins, ce texte n'apparaît pas répondre aux problèmes soulevés voire apparaît comme je disais tout à l'heure contreproductif pour lutter contre la récidive des violences conjugales. C'est notre travail de parlementaire. D'être sincère, écrire des textes pour écrire des textes, ce n'est pas la devise du Sénat. Ensemble soyons efficaces objectif pour protéger les plus vulnérables, que ça soit Madame Laborde Les femmes victimes mais aussi les enfants victimes et toutes les personnes vulnérables, nous avons encore beaucoup d'chose affermir. Madame Nicole Belloubet

Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur madame la sénatrice Laborde mais les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'initiative prise par le groupe RDSE et plus particulièrement par madame Françoise Laborde, que je voudrais ici saluer amicalement mérite toute notre attention, même si je le dis d'emblée le gouvernement ne pourra pas la suivre, pour des raisons que je développerai tout à l'heure, ces raisons d'ailleurs rejoignent pour l'essentiel celles qui celles qui viennent d'être exposé par Madame la rapporteure cette initiative que vous avez prises Madame la sénatrice Labor doit en effet être saluée car elle nous donne l'occasion de revenir sur la question des violences conjugales de ces violences inacceptables dont sont parfois témoins comme vous l'avez rappelé les enfants d'un coût de ces violences contre lesquels les pouvoirs publics mènent une politique qui est inscrite dans la durée, et ce avec une grande continuité d'action s'inspirant du régime qui est prévu par pour les auteurs d'infractions terroristes, vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, depuis la loi du 21 juillet 2016, le texte qui vous est soumis propose de durcir les conditions d'incarcération des auteurs d'infractions commises à l'encontre de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire de Pacs, plus précisément, ce texte prévoit en son article 1er que les personnes condamnées pour des faits de violence, de harcèlement d'enregistrement et de diffusion d'images violentes ou encore de viols commis à l'encontre de leurs conjoints ne pourront dorénavant plus bénéficier de certains aménagements de comme la suspension ou le fractionnement de peine de placement extérieur ou la semi-liberté, ce texte prévoit par ailleurs dans son second article que ces mêmes personnes ne pourront plus non plus bénéficier de crédits de réduction de peine, cette proposition a naturellement retenu l'attention du gouvernement tant celle de ma collègue, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes Madame Marlène Schiappa que la mienne, vous le savez, en effet, le ministère de la justice est particulièrement impliquée dans la lutte contre les violences conjugales, qui constitue l'une des priorités de la politique pénale, que nous portons et ce depuis de nombreuses années dans le même sens, j'attache également une attention toute particulière à la question de l'exécution des peines et de l'adaptation de notre politique pénitentiaire aux différents besoins de la société, ce sujet fera d'ailleurs l'objet d'ici l'été, de débat devant le Parlement dans le cadre de la loi de programmation pour la justice, qui comportera des mesures pénales pour redonner du sens et de l'efficacité à la peine, à cet égard, le gouvernement ne peut que se féliciter de l'attention portée par votre assemblée à ces questions, nous avons eu déjà l'occasion à plusieurs reprises en débattre tant au sein de la commission des lois que dans cet hémicycle, vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, je crois néanmoins que, si le texte qui nous est présentée aujourd'hui par d'un objectif louable, il pose des difficultés de principe, tant sur le plan juridique que d'un point de vue pratique les dispositions de la proposition qui est soumise, si elles étaient votées pour être ainsi et de manière paradoxale s'avérer plutôt contreproductive au regard de l'importante mobilisation dont fait actuellement preuve le ministère de la justice sur ces questions à travers une politique pénale et pénitentiaire méticuleusement construites ces dernières années pour ces raisons, donc je vous l'ai dit, le gouvernement ne pourra pas être favorable à ce texte, tout en n'en reconnaissant l'intérêt quant aux objectifs qu'il défend dans un 1er temps je souhaite donc évoquer les difficultés soulevées par cette proposition de loi, elles sont de 2 ordres : ce sont des difficultés d'opportunités et 2 constitutionnel en opportunité tout d'abord le mécanisme proposé exclut systématiquement les auteurs d'infractions commises sur leur conjoint de certains aménagements de or cette adaptation des modalités d'exécution des peines est indispensable en termes même d'efficacité, on le sait, et vous l'avez dit Madame la rapporteur, il n'y a rien de pire et vous-même d'ailleurs Madame la sénatrice, il n'y a rien de pire en matière de prévention de la récidive qu'une sortie sèche, une sortie de détention sans accompagnement par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ce que permettent justement les mesures d'aménagement de peine et en matière d'aménagement de peine, il convient, je crois, de laisser au juge d'application des peines, la plus large palette possible de mesures à sa disposition afin qu'il puisse mettre en place un suivi individualisé et adapté à la problématique de l'auteur, cette adaptation est en 1er lieu nécessaire car les faits de violences conjugales peuvent être extrêmement divers certains surviennent de manière habituelle au sein du couple, d'autres de manière ponctuelle, voire unique, par exemple dans le cadre d'une séparation en second lieu il n'y a pas, je crois, de profil type d'auteurs de violences conjugales, dans certains cas un contexte dépendance alcoolique chez l'auteur des faits peut-être détecté, il est alors impératif que que le juge d'application des peines puisse en tenir compte et qu'il aménage la peine afin de prévoir à cette occasion, une mesure de soins pour pallier cette addiction, cela peut permettre d'éviter de nouveaux passages à l'acte qui seraient liés à une telle addiction dans d'autres cas, les ressorts du passage à l'acte, peuvent trouver leurs racines dans une structuration pathologiques de la personnalité du caractère de l'auteur, quelle que soit cette structuration, on le voit, on ne peut donc en la matière, raisonner à l'aide d'un mécanisme prévoyant une exclusion automatique de telle ou telle mesure d'aménagement de peine les magistrats doivent resterait en mesure d'apprécier en fonction des faits commis des éléments de personnalité de l'auteur des expertises psychologiques qui sont réalisés du projet professionnel qui est présenté par le condamné de l'intérêt de la victime si l'octroi d'un aménagement est ou non opportun, j'insiste, à cet égard, sur le fait que la préservation des droits et la protection de la victime, font bien partie intégrante des critères examinés par les magistrats lorsqu'ils apprécient l'opportunité de l'octroi d'une mesure d'aménagement, ces ces mesures d'aménagement de peine que la proposition de loi qui vous est soumise, entend désormais prohibés pour ce type de condamner quelles sont telles qu'elles existent actuellement, il s'agit tout d'abord des mesures de suspension et de fractionnement de la peine, ces mesures peuvent être décidées pour motif d'ordre médical, familiale, professionnelle ou sociale et elles sont destinées à faire face à des situations particulières qui s'opposent, matériellement et en opportunité au maintien en détention les exclure pour une certaine catégorie d'auteurs d'infractions rendrait en pratique beaucoup plus complexe la prise en charge de ce public par l'administration pénitentiaire et par l'autorité judiciaire. Il s'agit ensuite de la semi-liberté du placement extérieur ces mesures permettent à l'heure actuelle, d'offrir un accompagnement et et un encadrement renforcé grâce à l'hébergement en centre pénitentiaire de semi-liberté ou bien dans une structure associative qui est conventionnée avec l'État en placement extérieur et je peux penser par exemple à l'association Emmaüs à l'Armée du Salut ou encore à l'association Horizon par exemple, de telles mesures s'certes également opportune lorsque sont prononcées dans ce cadre, certaines interdictions prévues par le code pénal, comme celle de résider hors du domicile conjugal ou de ne pas paraître à ses abords, elle permet également d'imposer à l'intéressé, certaines obligations, comme celle de fermer, objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, psychologique ou éducatives, enfin, il s'agit de la suppression des crédits de réduction de peine cette suppression des crédits de réduction de peine aurait des conséquences très négatives, me semble-t-il, sur la mobilisation des personnes détenues pour ce type de faits dans le cadre de leur parcours d'exécution de la peine, dès lors que leur mauvaise conduite en détention ne pourrait plus entraîner de retrait du crédit de réduction de peine par le juge d'application des peines si le dispositif que vous proposez, madame la sénatrice était adopté, il pourrait d'une certaine manière, et ce serait paradoxal en résulter un moins bon suivi en sortie des tensions, des auteurs de violences conjugales, par ailleurs, ces mêmes détenus pourraient ne plus être en cours encouragés à adopter un comportement adapté pendant la durée de l'emprisonnement à ces difficultés en opportunité s'ajoutent des difficultés de nature constitutionnelle, c'est le second point que je voudrais aborder et qui tient au fait que votre proposition se heurte donc je crois au principe constitutionnel vous le craigniez tout à l'heure, vous-même, la madame la sénatrice au principe constitutionnel d'égalité de de nécessité et de proportionnalité et d'individualisation des peines ces principes appliqués au cas présent existe en effet un traitement équivalent des auteurs d'infractions commises à l'encontre de leur conjoint vis-à-vis d'auteurs d'infractions de même gravité, or cette proposition de loi qui font d'un régime dérogatoire introduit une distinction qui est difficile à justifier endroits dans des situations de gravité équivalente, d'une part les condamnés visés par la proposition de loi se verront ont appliqué un régime plus rigoureuse que certains condamnés pour des infractions répliqué réprimer plus sévèrement par exemple une personne qui est condamné pour des faits d'agressions sexuelles commises sur un mineur de moins de 15 ans pourra bénéficier de l'ensemble des mesures d'aménagement de peine offerte par la loi, ainsi que de la totalité des crédits de réduction de peine, alors que la même personne condamnée pour des faits de violences par conjoint ne le pourra pas d'autre part, la proposition de loi ne vise pas toutes les infractions susceptibles d'être aggravées par la conjugalité mais seulement certaines d'entre elles, introduisant par là même une rupture d'égalité entre auteurs d'infractions au préjudice de leur conjoint ainsi à la lecture du texte proposé, il apparaît que le condamné pour violences conjugales sera exclu du bénéfice des crédits de réduction de peine et de certains aménagements, tandis que le condamné pour agression sexuelle sur son conjoint pourra quant à lui en bénéficier pour ces raisons, l'avis du gouvernement concernant cette proposition de loi défavorable pour autant l'occasion m'est donnée d'insister sur les actions que nous menons en la matière et je tiens à vous assurer, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs que sur le fond, nous rejoignons pleinement les objectifs poursuivis par la proposition de loi visant à mieux protéger les victimes de ce type de faits qui sont tout à fait inacceptable ainsi après avoir évoqué les difficultés soulevées par la proposition de loi je voudrais brièvement rappelé les dispositions légales en vigueur qui permettent déjà me semble-t-il, une prise en charge efficiente des auteurs de ces infractions, le ministère de la justice dans l'autorité judiciaire et que l'administration pénitentiaire, même temps, en effet, en la matière. Une politique pénale et pénitentiaire particulièrement volontariste visant tout à la fois à prévenir la récidive chez les personnes condamnées mais également à mieux protéger les victimes. En matière de prévention de la récidive dans le cadre du suivi des personnes placées sous main de justice, les services d'insertion et de probation mettent en oeuvre sous le contrôle du juge d'application des peines, des modalités de suivi individualisé et différenciée en fonction des problématiques à l'origine du passage à l'acte délictueux les méthodes utilisées, qu'il s'agisse d'entretien motivation de groupes de parole Vista modifier les schémas comportementaux des personnes condamnées pour violences conjugales en les sensibilisant à la question de l'égalité femmes-hommes, à ce titre, plusieurs dispositifs spécifiques sont mises en oeuvre par l'administration pénitentiaire, en lien notamment avec les associations spécialisées, et plus particulièrement avec celle qui interviennent en matière d'aide aux victimes ainsi en milieu fermé des actions visant à lutter contre les stéréotypes fondés sur le sexe dans les lieux, privation de liberté sont mises en place dans ce cadre, on veille à ce que la gamme des formations ou des activités proposées aux personnes détenues y compris qui les activités sportives et culturelles, souhaite aussi large que possible l'ennui en y incluant des dimensions liées au respect d'autrui aux violences conjugales et aux violences faites aux femmes. En milieu ouvert et en milieu fermé, les services d'insertion et de probation développe des dispositifs de prise en charge collective sous la forme de groupes de parole, animé par des conseillers d'insertion et de probation appelé programme de prévention de la récidive ces programmes Vista faire travailler collectivement les condamnés sur le passage à l'acte délictueux et sur ses conséquences pour la victime et pour la société, il est ainsi question de confronter les vécus et d'apporter un certain nombre de repères, rappel à la loi, éducation civique mise en commun des expériences à des détenus ou à des probation ayant commis des actes de même nature afin de faire évoluer la représentation que se font les intéressés, de leur geste et ainsi de prévenir la réitération du passage à l'acte en 2016, 35 programmes de prévention de la récidive relatives aux violences conjugales et intra-ont ont ainsi été organisées sur le territoire national, au bénéfice de 1360 personnes placées sous main de justice cette démarche dynamique de prévention de la réitération de la récidive trouve également une illustration à travers le développement en milieu ouvert, des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences au sein du couple et sexiste. Stage créé par la loi du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en 2016 67 stage de cette nature ont été organisées au bénéfice de 388 personnes placées sous main de justice. En matière de protection des victimes également nous accomplissons un certain nombre d'actions pour protéger les victimes de violences conjugales en complément des dispositifs juridiques déjà existants, permettant notamment l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, le ministère de la justice généralise actuellement un dispositif qui a fait ses preuves, le téléphone grave danger ce ce dispositif de télé protection peut-être attribué pour une durée de 6 mois renouvelable par le procureur de la République à une victime de violences conjugales dont l'auteur est soumis à une mesure d'interdiction d'entrer en contact, ce dispositif est d'une grande utilité pour sécuriser les femmes victimes de violences conjugales, le TGD puisque c'est le nom de ce téléphone grave danger le TGD permettent en effet d'alerter rapidement les forces de l'ordre et de géolocaliser la personne bénéficiaire si celles-ci sont en danger en décembre 2017 543 TGD étaient déployés en juridiction, mais dans le cadre d'un nouveau marché public, entré en vigueur en 2018 le nombre de TGD sera prochainement porté à 634, Tél ce ce déploiement du TGV s'inscrit dans le cadre du nouveau plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes, pour la période 2017, 2019 qui prévoit de nombreuses mesures parmi lesquelles le déploiement du dispositif TGD dans les départements d'outre-mer,

est d'une politique publique particulièrement volontaire et abouti qui s'inscrit dans une grande continuité d'action je tiens ici à le redire depuis plusieurs années, je voulais vraiment le souligner les peines encourues en matière de violence conjugale, qui je vous le rappelle, sont de 3 à 10 années d'emprisonnement en fonction de l'incapacité totale de travail constatée cette peine en matière de violence conjugale et la politique pénale qui est empreinte de fermeté menées par les parquets attestent de la pleine conscience et de la mobilisation des pouvoirs publics dans la lutte contre ce type de faits tout simplement inacceptable ne peut toutefois se réduire à une approche purement sécuritaire et un traitement qu'on pourrait qualifier de d'exclusivement carcéral des auteurs de ce type de faits à travers la politique pénale et pénitentiaire que je viens de décrire le gouvernement souhaite consolider l'édifice patiemment et méticuleusement méticuleusement construit tout au long de ces dernières années, afin de prévenir les violences conjugales, de protéger les victimes et de réprimer les auteurs pour l'ensemble de ces motifs et malgré tout l'intérêt que présente cette proposition le gouvernement ne pourra que donner un avis défavorable au texte qui nous est proposé, vous remercie. Merci alors pour que vous soyez tous dans la maîtrise de 7 heures du jour avec l'ensemble des connaissances que vous de donner Si nous poursuivons la discussion générale, jusqu'au bout avec les inscrits et leur temps de parole nous dépassons de plus de 10 minutes le temps limite de cette ce qui m'était impossible selon les consignes que je reçois, on peut dépasser d'une 2 minutes pas du 10 donc je vous propose la chose suivante, c'est que chacun par solidarité essaye de réduire un petit peu et nous allons peut-être y arriver aussi non, les 2 derniers ne pourront pas intervenir. Parce que la discussion sera Close et quand je dis les 2 derniers, c'est un peu plus mais on va dire les 2 derniers, pour l'instant. Donc voilà, tout ça est entre vos mains, si chacun lâché une petite minute dans son intervention va peut-être y arriver monsieur Roland Courteau à la parole, pour 5 minutes. C'est le président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission Madame le rapporteur, on aurait pu croire en ce début du 21ème siècle que les violences conjugales, ce mal, d'un autre âge ne serait aujourd'hui que très lointaine et très mauvais souvenir et il y a appartenu à un lointain passé, mais il n'en est rien, hélas c'est insupportable fléau d'toujours pas de faire des ravages Hollande pas sous-estimé minimisé, il est resté trop longtemps tabou, il est vrai que le meilleur moyen de s'accommoder d'un mal qui dérangeait, c'était à l'époque de l'ignorer, d'où ma première proposition de loi que j'ai souhaité porter ici même, lave, mars 2005 et qui la loi du 4 avril 2006 loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple cette première loi spécifique a amorcer un mouvement qui je crois ne cessera pas et qui va dire, a été prolongé par plusieurs autres lois plusieurs plans et mesures diverses et par nombre de d'initiative de la part notamment de Laurence Rossignol que que je salue au passage en sa qualité de ministre et puis merci aussi à vous, madame la ministre de la justice de votre implication sur ce dossier particulièrement sensible, je salue à ce stade de mon propos également votre joint Costa Amflora Françoise Françoise Laborde à lutter contre ce fléau, mais comme vous le soulignez, malgré toutes ces dispositions des violences conjugales, demeure une triste et inacceptable réalité face à ce constat, vous proposez de modifier de manière drastique le régime de l'exécution des peines, des auteurs de violence des peines qui déjà dans cette loi de 2006 fortement aggravée pour les faits de violence commis au sein des couples. De plus, la loi de 2010 à renforcer les sanctions avec l'aggravation des peines en cas de menaces proférées au sein du couple, y compris dans le cas d'Elior lasse psychologique ou de harcèlement moral, bref les peines encourues sont déjà considérablement, ce qui paraît légitime par rapport à des comportements destructeurs, faut-il alors aller plus loin encore, je comprends votre colère Françoise Laborde quand vous dénoncez dans votre texte le décalage entre la réalité du drame vécu par les victimes et leurs familles et la priorité donnée dans le débat public à la lutte contre les violences faites enfin je comprends d'autant mieux et action qu'il a pu arriver que des auteurs de violence était DC en liberté. D'où la réaction des familles et des victimes que je comprends parfaitement, toutefois, nous ne pensons pas avec le groupe socialiste pouvoir vous suivre cette fois-ci sous certaines des dispositions que vous proposez dans ce texte, ainsi est-il proposé d'exclure du bénéfice de fond du fractionnement ou de la suspension de la peine, les personnes condamnées pour violences au sein du couple je note d'abord que plusieurs des infractions ciblées étant de nature criminelle leurs auteurs ne peuvent déjà pas bénéficier de ces aménagements, quant aux intentions en correctionnelle lisez-il comme il a de l'autre et dans ce cas, cas, le juge de l'application des peines peut déjà refuser telle ou telle aménagement puisque le condamné doit remplir un certain nombre de conditions pour en bénéficier, même remarque concernant la proposition de ce cuir du bénéfice du régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, les personnes condamnées pour ces mêmes infractions, de l'application des peines, l'opportunité de juger selon les cas, sans oublier que la semi-liberté prépare à la réinsertion et peut prévenir la récidive à ce sujet, je voudrais rappeler ce sur quoi j'avais beaucoup insisté lors de l'examen de ma première proposition de loi, je veux parler de la prise en charge sanitaire, social ou psychologique et donc de la nécessité pour le condamner de suivre, je cite, une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, c'est d'ailleurs l'un des 3 critères pouvant justifier une réduction supplémentaire de peine mais qu'il s'agisse d'exclure les réductions de peine ou les réductions supplémentaires de plaine, prenons garde à l'effet l'effet productif de la mesure, si le code n'sait par avance qu'il en est écarté et je doute qu'ils soient incités à suivre régulièrement et sérieusement des swing qui serait à même de réduire au maximum les risques de récidive, je comprend vos préoccupations Françoise Laborde mais il semble préférable, pour des raisons que je viens des mots clés puisque l'arsenal législatif est déjà sévère à l'encontre des auteurs de violence, d'axer nos efforts en direction des recommandations que nous avons mise en avant d'un autre rapport au nom de la délégation aux droits des femmes rapport intitulé violences conjugales un combat inachevé, je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues. Une femme meurt tous les 3 jours sur les coups de son compagnon ou son ex-conjoint. Malheureusement, ce chiffre ne reflète pas l'arrêter, car il n'intègre pas les données concernant les consécutifs Obiang psychique et psychologique ainsi que ce qu'elle a engendrée par la console psychotropes de tabac ou d'alcool. En 2016, 110000 victimes de violences commises par leur conjoint, concubin ou est-ce conjoints ont déposé plainte auprès des services de police entraînera la condamnation de seulement 17 ni sur une personne pour violence conjugale.

Cette proposition de loi part du constat, les énormément de peine et cris de réduction de peine entraîne un sentiment d'impunité pour les auteurs, auteur de ces violences et un sédiment d'incompréhension et d'montant pour les victimes et leurs proches. Ce texte en temps assis à prévoir la création d'un régime dérogatoire afin notamment de mettre un terme à la non-exécution de petites peines donc raisonnement lorsqu'elle révèle de ces faits toutefois cette profession de loi appelle à forme de remarques. Tout d'abord concernant et infractions retenues pour la vous article celle celui-ci recouvre des viandes inégale gravité en excluant l'homicide et en incluant le harcèlement téléphonique ou le harcèlement moral au travail en outre certaines infractions pénales, il y a notamment à la répression des violences faites en groupe ne peuvent pas être commises à l'encontre d'une victime par son conjoint ou compagnon. Ensuite, article 1er aurait pour conséquence d'empêcher le prononcé de sa mesure probatoire encadrant les sorties de détention comme des mesures de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, alors que celle-ci pourrait permettre de réduire le risque de récidive enfin aussi l'article 2 qui prévoit la création d'un régime dérogatoire pour les auteurs de violences conjugales 7bis position porterait inévitablement atteinte aux principes essentiels devant la loi. Au cours de l'examen de ce texte en commission des lois.

d'aménager Attigny bio au stade du jugement, les peines d'emprisonnement prononcées, d'une durée inférieure ou égale à 2 ans ou pour le juge d'application des peines de prononcer une mesure de placement sûr séquences électroniques, elle a également rappelé je qu'Al-Qaïda d'options en en octobre 17 de la proposition de loi d'orientation et de programmation peut redressement de la justice, la commission des lois, avait déjà proposé une réforme d'envergure du régime exception des peines. Même si des progrès substantiels doivent être accompli de nombreuses avancées ont été réalisées en matière de protection civile et pénale des victimes de ces violences depuis 1994 les peines encourues par les eaux turbulences conjugales sont aggravées lorsqu'on a lorsqu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin cette circonstance aggravante est élargie aux partenaires liés à la victime par un Pacs, ainsi qu'à son ancien conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs par la loi du 4 avril 2006 qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, enfin, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce le droit civil organise également l'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile commun, en effet, lorsque celle-ci exercée par l'un des époux mettent en danger son conjoint et. et. Un ou plusieurs enfants, le juge d'affaire Pagnol statue en amont de la poussière de divorce sur la résidence séparée des époux une mesure d'éviction peut également être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire depuis le 5 mars 2007 on a-t-il un pensionnat la délinquance, les personnes reconnues coupables lance conjugales peuvent également être condamné à ainsi socio-judiciaire en complément, une ordonnance de protection de ses victimes peut également être délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales depuis la loi du 9 juillet 2010, le juge pas leur retirer l'autorité parentale au parent condamnés comme auteurs ou complices d'un Crime sur l'autre parent,

Madame la Ministre, mes chers collègues, je partage pleinement l'objectif poursuivi par l'auteur de la position de loi, c'est-à-dire l'amélioration de la lutte contre la violence conjugale, néanmoins je regrette que ce texte soulève trop de juridique et pratiques pour être adopté ainsi pour toutes ces raisons, le groupe les indépendants ne votera pas en faveur de cette loi. la parole est à monsieur Guillaume Armelle. Pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre Madame la rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs, mais, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui porte sur un sujet d'importance qu'ils méritent, on flotte attention et surtout toute notre implication, je souhaite pour ma part félicitées ma collègue François ce qu'il y a en a pris toute la mesure et nous propose une modification de notre législation mais, chers collègues, la violence conjugale est un vrai fléau encore trop présent dans nos sociétés, qui tous les 2 7, il faut le rappeler, même si les victimes sont principalement et de très loin les femmes, le rapport du Conseil économique, social et environnemental intitulée Combattre les violences faites aux femmes dans les outre- mer révèle que sur l'ensemble du sol national, 88 pourcent les fuites futiles des violences conjugales sont des femmes et 80 6 pourcent des violences sexuelles sont subies par les femmes, il s'agit bien entendu et destination a minima, puisqu'il est impossible de recenser toutes les violences non dentelle ne faisant pas l'objet de poursuites, mais vous en conviendrez avec moi mais, chers collègues, ces chiffres sont affolants le même rapport précise également que ces violences faites aux femmes sont une des conséquences des stéréotypes ancrés dans toutes les sociétés assignant les hommes et les femmes à des rôles de sexe et à des rapports de domination des hommes sur les femmes, il s'agit donc de phénomène culturel, entre guillemets, très ancrée dans nos sociétés et il faudra encore beaucoup de temps avant de l'éradiquer totalement, mais plutôt nous nous y attaquons, plus vite nous y parviendrons en moins de ultramarins je n'oublie pas la situation des outre-mer qui est encore à bien des égards beaucoup plus affolantes, je me rappelle de l'intervention de ma collègue, on connaît ici même à la tribune, le rapport d'Ernestine Ronai, pour le compte du CESE que je citais précédemment souligne que la situation, les territoires ultramarins n'est pas uniforme l'insularité, la faible superficie des certains territoires peuvent entraver la libération de la parole des victimes ébranle l'inopérant l'éloignement de la personne violant le travail d'éveil des consciences ne peut donc pas s'effectuer de la même à la même vitesse et de la même façon sur l'ensemble du territoire s'il est possible de mette fin à ces violences, du jour au lendemain, il est absolument nécessaire que le gouvernement poursuive et intensifie les politiques publiques ciblée sur cette problématique en ayant une approche spécifique pour les territoires ultramarins l'objet un notre débat aujourd'hui ne porte pas sur les violences conjugales en elle-même mais plus spécifiquement sur le régime de l'exécution des peines des auteurs des violences conjugales, cependant il me semblait opportun et important de rappeler, c'est une réalité bien qu'améliorée par l'arrêt de l'éviction du conjoint violent du domicile, la mise en sécurité des victimes reste un parcours long et complexe qui se prolonge parfois après la condamnation judiciaire de l'auteur des violences, mais la situation actuelle n'est pas satisfaisante à bien des égards les fréquences d'aménagements de peine, peuvent entraîner un sentiment de grande incompréhension chez les victimes et leurs familles quand il ne les mettent pas en danger directement plus largement ces aménagements de peines peuvent substituer suscité pardon l'incompréhension de ce qu'il croit ce qu'qui voient une disproportion entre la gravité des faits reprochés et la peine effectuée par le coupable, j'y vois pour ma part 2 conséquences : d'une part cela peut décourager les potentielles victimes de porter plainte contre leurs bourreaux de peur de lui voir celui-ci se venger et, d'autre part, les peines et leurs aménagements ne sont absolument pas dissuasif pour les auteurs des violences conjugales pour remédier à ces phénomènes, la présente proposition de loi et nous en sommes conscients n'apportera pas toutes les réponses, mais propose de modifier l'origine de l'exécution des peines, des auteurs de violences conjugales, afin de les maintenir à une distance effective de leurs victimes, les membres de la commission des lois, ont estimé que le texte n'était pas acceptable en l'état et nous comprenons livraison, il ne sera peut-être pas adopter ou sûrement pas adopté par nos trois-quarts mais il nous plairait fortement Madame la Ministre, que le gouvernement s'engage à se saisir de cette question spécifique du régime de l'exécution des peines, les auteurs de violences conjugales dans sa globalité mais aussi en tenant compte Merci. La parole est à monsieur Thani Mohamed pour 6 minutes aussi la République en marche. Président Madame la Ministre, mes chers collègues, dans notre pays en 2016, 157 personnes ont trouvé la mort, victime de violences de leur partenaire ou ex-partenaire 78 pourcent de sa fuite de ses victimes étaient des femmes. Dans les plaintes déposées pour coups et blessures volontaires de la part de conjoint ou ex-conjoint 87 pourcent des femmes étaient également des victimes en 2016, il est important de préciser que nous sommes probablement très en deçà de la réalité car les enquêtes de victimation, ont montré que seuls 14 pourcent des victimes de violences conjugales déposent plainte, la prévalence du nombre de femmes touchés et l'augmentation du nombre de victimes de violences conjugales chaque année est une constante

d'agressions physiques contre les femmes ont été constatés, selon ces chiffres jusqu'à 8 fois plus d'agressions sexuelles par conjoint ont également été constatés au-delà de de ces chiffres, ce sont des drames souvent familiaux qui se joue, comme l'actualité la tristement rappelé ces derniers temps, il s'agit d'un sujet éminemment sensible et la lutte contre les violences conjugales, largement partagée, cependant, cette proposition de loi qui qui a le mérite d'avoir porté, encore une fois ici ce sujet très ça très sensible, mon groupe ne peut pas y souscrire pour les raisons qui ont été rappelé tout à l'heure que je, je, je, je rappelle, avec le temps, raccourci les raisons d'hostilité, je suis hostile aux lois d'exception qui ne prennent en compte ni le principe de proportionnalité, ni celui d'individualisation des peines pour les raisons de contre-productivité pour prévenir les récidives qui ont été avancés tout-à-l'heure par Madame la rapporteur pas madame la garde des Sceaux également et puis aussi pour la raison suivante, c'est que les les dispositions qui sont prévues par cette proposition de loi pourrait avoir pour conséquence d'inciter les juges à prononcer des peines plus faible pour prévenir, pour prévoir, pardon, des aménagements à Benicio et vous en conviendrez Madame ça serait l'effet inverse recherché par votre proposition de loi, enfin la la raison d'inconstitutionnalité celle-là et les également importante, la dénonciation des violences conjugales reste encore un sujet tabou dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de de circonstance, je crains que la solution pour lutter contre ce type de violence se trouve moins dans le durcissement du régime des peines que dans l'amélioration de l'application du droit existant et la prévention il convient surtout d'oeuvrer à renforcer la protection des victimes et à délier les langues pour toutes ces ces raisons, et malgré la pertinence et l'acuité de votre peine, chers collègues, nous ne pouvons pas la soutenir en l'état. Merci Madame Éliane Assassi. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologistes Merci monsieur le président Touré Dabo remercier de m'avoir permis de prendre la parole ce soir en raccourcissant ses propos Madame la miss mis chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui par nos collègues du groupe RDSE aborde donc un sujet très sensible et s'inscrit dans un contexte très préoccupant en 2016 2016 123 femmes et 34 hommes ont été tuées par leur conjoint ou leur conjointe, en moyenne, donc 225000 femmes par an sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur anciens ou actuels partenaires, ces chiffres sont effrayants mais plus effrayant encore moins d'une femme sur 5 victimes de violences conjugales porte plainte, loin de s'attaquer à cette question précise de la libération de la parole et surtout du recueil de celle-ci, la proposition de loi de Madame Laborde se concentre sur l'exécution des peines, des auteurs de violences conjugales de violences conjugales, je ne reviens pas sur les contenus des 2 articles proposés, bien évidemment, les intentions de Madame Laborde sont louables mais dire dans l'exposé des motifs que ces aménagements de peine laisse installer un sentiment d'impunité pour l'auteur de ces violences n'est pas à la hauteur de l'enjeu et s'inscrit dans une logique qui peut être contre-productif, dans l'approche de tout sucé, sujet sensible qui soulève une émotion bien légitime chez nos concitoyens, je pense qu'il est de votre devoir de garder la hauteur d'esprit qui s'impose et surtout de préserver les valeurs de notre République et l'équilibre de notre droit, nous partageons une bonne partie du diagnostic de madame la rapporteure quant aux mesures à approuvé proposer et donc Johnny on vient pas mais je veux simplement insister sur un aspect car cette proposition de loi apparaît porteuse de rupture d'égalité devant la loi, c'est en effet le quantum de la peine trop non et le prononcer ou non d'un mandat dépôt qui détermine les modalités d'exécution d'une décision de condamnation, celle-ci de dépendent pas simplement de la nature de l'instant infractions visées mais prennent en compte la gravité des faits et la personnalité de l'auteur, finalement, l'État les dispositions qui nous sont proposées peuvent fragiliser l'équilibre de notre droit pénal, puisqu'elle porte atteinte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi de nez Cissé de nécessité de proportionnalité et d'individualisation des peines, c'est en ce sens que les membres du groupe communiste républicain et citoyen écologistes s'étaient déjà opposés au régime de l'exécution des peines dérogatoire applicable à certains condamnés pour une infraction peu à peu des régimes juridiques d'exception s'installe avec des droits spéciaux hier pour les terroristes aujourd'hui pour les auteurs de violences Conche conjugal et demain, pour qui, mais, chers collègues, revenons aux fondamentaux ne confondons pas justice et vengeance en matière de droit pénal, bien loin de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice de Monsieur bah, à laquelle se réfère la rapporteure, nous réaffirmons la nécessité d'une réflexion d'ampleur à la fois sur l'échelle et le sens de la peine qui éviterait ce genre de débat qui, pourtant, je le répète, à bord d'une question de société primordial, mais rappelons que les situations de violences conjugales relève d'abord majoritairement de situation d'impunité dans leur très grande majorité des violences conjugales n'arrive jamais devant la justice, je le redis, moins d'une femme sur 5 victimes de violences conjugales porte plainte, c'est donc d'abord à cette impunité qu'il faut s'atteler, en renforçant les moyens que ce soit pour les policiers, qui accueille les victimes et reçoivent les plaintes ou pour les juges et la justice, de manière générale, en outre, les conditions doivent être créées pour que la loi et les avancées qu'elle a déjà permis soient réellement appliquée éviction du conjoint violent, téléphones portables, donc j'ai médiation pénale, d'autres avancées sont encore possibles, je pense, notamment, madame la ministre, à la création de nouveaux hébergements d'urgence, en élargissant, en élargissant ce qui se fait déjà en terme de conventions avec des offices HLM dans certains départements, conclusion, ce sont ces solutions que nous affirmerons et que 12 à fileront et réaffirmerons dans les mois à venir, notamment lors des discussions, des projets de loi de la chancellerie et du secrétariat d'aide à d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes qui au soulèveront la question des violences faites aux femmes à ces occasions, nous ne manquons pas de veiller à ce que la question soit traitée dans sa globalité, dans le respect de l'équilibre de notre droit, et non sous l'angle de la surenchère répressive. je vous remercie Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur madame l'auteur les chiffres des violences conjugales dépeignent situation alarmante en 2016 plus de 120000 femmes ont subi des violences et 123 sont mortes sous les coups de leur conjoint, la lutte contre les violences conjugales est donc loin d'être achevée, ce qu'il appelle en amont à la prévention de tels actes et nécessitant en aval de réfléchir à la sécurité des victimes, en particulier après la condamnation judiciaire du conjoint et sa libération. Engager une réflexion sur notre régime des écussons des peines comme le propose le la présente proposition de loi paraissait tout à fait légitime. Le présent texte vise à créer un régime dérogatoire en matière d'aménagement des peines applicables aux seuls auteurs de violences conjugales, ces derniers seraient ainsi exclus de la plupart des possibilités d'aménagement de peine : nous sommes et chers collègues, face à un sujet éminemment sensible, mais il est essentiel d'aborder ce débat avec raison. Et rigueur juridique afin que nos décisions permettent d'apporter un réel soutien au vu. C'est dans la discussion précédente, nous évoquions les risques. D'une loi mal écrites, qui risquent de provoquer des effets qui ne sont pas ceux qui sont attendus, or si nous comprenons et partageons l'objectif de ce texte afficher davantage de fermeté vis-à-vis des auteurs de violences conjugales, nous regrettons que son contenu soit inapte à atteindre cet objectif, pire, nous craignons je viens de le dire, qu'il soit contre-productif privé les personnes condamnées pour violences conjugales, de la possibilité de bénéficier d'un aménagement de peine, c'est méconnaître l'objectif 1er des peines restrictive et privative de liberté à savoir préparer les personnes condamnées à leur propre réinsertion dans la société, il ne s'agit pas de considérer ces aménagements uniquement à l'aune des avantages qu'il représente pour la personne condamnée mais de prendre aussi en compte tous les bénéfices que notre société en tire notamment en termes de prévention de la récidive sur ce plan la présente proposition de loi semble ignorer que le lien de causalité entre ce qu'on appelle les sorties sèches et la récidive de longue date, été établi par ailleurs qu'il est important de rappeler que des aménagements de peine, comme le régime de semi-liberté ou le placement à l'extérieur, permettent de concilier protection des victimes et prise en charge de la personne condamnée aussi ce texte voté louable dans ses intentions, attention, nous pouvons partager une empreinte malheureusement pas, selon nous, la bonne direction, il y aura toutefois permis d'ouvrir la voie à une indispensable réflexion sur la lutte contre les violences conjugales et l'eau permettant avait déjà préparé la discussion du futur projet de loi que portera madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la perspective de ce débat, il faudra garder à l'esprit que la lutte contre les violences conjugales ne doit pas être exclusivement abordé sous l'angle des sanctions pénales contre leurs auteurs en effet l'ampleur judiciaire de ce phénomène n'est pas à la mesure de sa réalité quotidienne aujourd'hui, seule une femme victime de violences conjugales sur 5 porte plainte, les sanctions ne concerne donc qu'une infime partie des infractions réellement commises la parole se libère 7 heures, cette situation est intolérable et il nous faudra trouver des solutions pour libérer vraiment dans notre société cette parole qui était c'est par peur des représailles, nous sommes dans le cadre de la famille et c'est souvent une difficulté, l'acteur de se rendre au commissariat pour déposer une plainte n'est par ailleurs ni simple ni aisé pour aucune des femmes qui doit le l'accomplir et cette étape constitue une épreuve supplémentaire pour nombre de victimes qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer ou craignent dit être mal accueillis par des personnels, souvent peu formés à cet exercice : ouverture d'une plateforme de signalement en ligne pour les victimes de violences, annoncé en novembre dernier, marquerait pour les victimes, un réel progrès et permettrait de rendre leur parole audible mais chers collègues. Le groupe de l'Union centriste, votera contre cette proposition de loi, au vu des insuffisances précédemment évoqués, et si nous nous inscrivons dans la volupté tout du président de la République de voir qui a fait de cette question de l'égalité de, de, de toutes ces questions-là, la priorité de son quinquennat nous espérons que les débats que nous aurons sur ce sujet à l'avenir, nous conduirons adopter des mesures aptes à lutter efficacement contre les violences conjugales, un message fort qui seraient envoyés aux victimes de ces violences et c'est surtout le nombre de ses victimes que nous pourrions enfin faire diminuer dans notre pays. Merci. Quand même souligner alors monsieur PELE va va monter pour parler. Que cet hémicycle fait preuve de grande solidarité puisque nous avons récupéré 9 minutes 30 pour que les 2 derniers puisse parler, bravo à vous. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois Madame le rapporteur, mes chers collègues, les violences conjugales sont un fléau contre lequel nous devons nous lier, hommes et femmes afin de combattre les chiffre sont criants, ils ont été largement rappelée, mais Jean mentionnerait de de 3 femmes, victimes sur 4 4 déclare avoir subi des faits répétés 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales, c'est trop, la proposition de loi de notre collègue Françoise Laborde visant à modifier le régime de l'exécution des peines, des auteurs de violences conjugales, propose d'empêcher les conjoints, concubins, partenaires des victimes de violences conjugales, de bénéficier de la suspension ou du fractionnement de paiement qui peut être autorisée par le juge pour motif odeur médicale, familiale, professionnelle ou sociale prévue à l'article 720 26 rien du Code de procédure pénale de l'exécution de la peine en semi-liberté ou en placement à l'extérieur, prévue à l'article 723 tirer un du Code de procédure pénale du bénéfice des crédits de réduction de peine prévue à l'article 721 du code de procédure pénale, le souhait de les exclure de ce dispositif afin de les maintenir à distance effective des victimes le plus longtemps possible à titre personnel, je comprends, et vous n'avez pas eu besoin de me convaincre, Madame la sénatrice n'aborde de l'intention de la proposition de loi, néanmoins, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une solution valable sur la forme, je ne nie pas l'angoisse des victimes mais retardé toutes sortir en interdisant réduction et aménagement de peine ne leur apportera rien ses auteurs de violences conjugales incarcéré finiront tôt tout tard par sortir de prison et de ne plus avoir, mais d'une plus sans avoir eu le moindre suivi, or nous connaissons l'utilité des aménagements de peines qui sont constitués de suie probatoire dédié de traitement et d'obligation de soins, je crains que les priver de ces dispositifs ne soient pas favorables à la lutte contre la récidive. Le régime des aménagements de peine ne doit pas être remis en cause et s'il était, pour les auteurs de violences conjugales, nous ouvrions la boîte de Pandore car il devrait l'être dans de nombreux autres situations. Cette proposition de loi fait face à un autre obstacle est un obstacle de taille, ce régime dérogatoire en matière d'exécution des peines qui serait applicable aux seuls auteurs de violences conjugales est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, nous touchons là à la constitutionnalité du texte. Vous l'aurez compris gel ou l'intention de la proposition de loi mais il est impossible de la soutenir au vu des raisons que j'ai évoqué le droit positif peut certes être améliorée, mais nous devons trouver d'autres voies, l'intérêt de ce texte et surtout d'ouvrir le débat et je remercie l'auteur Françoise Laborde, vice-présidente de la délégation droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes de l'avoir entrepris toutes les pistes doivent être envisagées, un autre plan que celui de l'exécution des peines doit notamment être améliorée, nous devons veiller au droit de la à la formation des victimes, il faut qu'elle soit informé de la date précise et les conditions de sortie de leurs agresseurs, c'est ce qui ressort de certains forums autre voie à suivre l'éducation dès le plus jeune de plus jeune âge à la lutte contre les violences envers les femmes à ce titre, la Fondation UFA pour l'enfance a par exemple financé et aidé à développer un programme dénommé de ce qui a prouvé son efficacité en Inde et en Océanie, les chiffres dans le Pacifique sont consternants des femmes ont déjà été battus par leurs partenaires et 75 pourcent des adolescents garçons interroges estiment qu'il est acceptable de frapper sa femme le programme Jospeh enseigne aux jeunes du Pacifique à travers le foot, le respect, la tolérance entre les 2 sexes, les résultats sont probants les mentalités de ces jeunes depuis son introduction en 2009 ont changé apprendre des la de l'essence, l'égalité des sexes et sensibiliser à la lutte contre la violence conjugale pourrait être une voie intéressante et peu onéreuse. Avant de conclure : je souhaite remercier Madame le rapporteur Brigitte Lherbier pour la qualité de son travail et dans cet important dossier relatif aux violences conjugales je tiens encourager vos travaux, madame Lagarde Esso et se de, de Madame, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femme enfin j'aimerais citer les travaux de la délégation entre les femmes et l'égalité homme femme dont j'étais vice-président durant ces 3 dernières années et qui fait un énorme travail d'audition d'analyse, de réflexion sur la vie de sa présidence, Annick Billon, je vous remercie pour être attention. merci, la parole monsieur Jacques Bigot, là je vais être plus directif pour que les 2 derniers interviennent, c'est-à-dire monsieur Laménie derrière, au lieu d'avoir chacun 5 minutes leur propose d'en avoir 3 et demi chacun.

tout a été dit sur le sujet, d'abord sur l'importance du sujet aussi sur la l'impossibilité dans laquelle nous sommes de de voter, je voudrais vous remercier, Madame la ministre d'avoir très objectivement et de manière très complète démontrer tout ce qui se mettent en je merci Roland Courteau d'avoir rappelé le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir et ce chemin-là, c'est essentiellement comme d'autres l'ont dit la nécessité surtout de sensibiliser les femmes parfois aussi désormais essentiellement des femmes à porter plainte et à ne pas se laisser faire et c'est cela qui est important et ce n'est pas la sanction pénale qui aboutira, ce sont les poursuites, ce sont les informations, c'est les travaux qui ont été faits depuis des années par des associations qui ont accompagné les femmes victimes qui ont permis de se soustraire du domicile conjugal, etc, mais ce texte doit être aussi l'occasion pour nous de dire ce que doit être une sanction pénale, elle a d'abord une première mission c'est sanctionné un manquement à l'ordre public et on est clair, que des violences intrafamiliales sont une atteinte à l'ordre public, elle doit ensuite permettre la réinsertion de la personne parce qu'on sait très bien que la personne délinquante ne restera pas indéfiniment en détention et enfin doit protéger elle très FICA, c'est protéger la victime, ce qui est dans ce domaine-là particulièrement important mais cette protection, elle ne peut se faire que si l'on donne aux juges, que ce soit le juge d'application des peines, le juge correctionnel ou la Cour d'assise ou le juge aux affaires familiales, les moyens de s'adapter à la nécessité particulière de ce service et donc sur ce sujet : nous avons raison d'en parler publiquement, mais nous devons être extrêmement sur le contenu de la loi, nous devons donner les outils et les moyens financiers de faire et je me souviens, madame la garde des Sceaux de la manière dont ont été mis en place les premiers téléphones à Strasbourg, le procureur de la République avait obtenu du président de la communauté urbaine que j'étais à l'époque que nous financiers ont, sur les 2 minutes le le téléphone et ça a été une expérience efficace et dans combien de départements, ce sont les départements qui, au titre de l'action sociale sont intervenus donc nous voyons bien que la justice aura besoin non pas d'une loi Madame Laborde mais de moyens financiers pour faire face à ce défi, la justice et la miss ration pénitentiaire, je le rappelle. Merci Monsieur Bigot monsieur Marc Laménie, vous avez la parole. Oui merci monsieur le président, Mesdames, la garde des Sceaux, c'est le président de la commission des lois, âme reporters chers collègues et puis merci de la solidarité et je crois que dans cette proposition de loi, je crois que c'est la notion de solidarité, de prise de conscience et merci Françoise Laborde et ses collègues du groupe RDSE d'avoir abordé un sujet extrêmement sensible concernant cette proposition de loi en rappelant cette prise de conscience indispensable je rappellerai aussi bah tout le travail qui est fait au niveau de la délégation de devront défendent présidée par notre collègue Annick Billon, sujet de société très sensible, je crois que c'était vraiment rappeler sur par l'ensemble de tous les intervenants, rappelons aussi le travail de la commission des lois, parce que je crois que c'est aussi très très sensible l'implication du ministère de la justice, vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, ont redonné le sens et l'efficacité dans le cas de l'exécution des peines cependant sur été rappelé les faits de violences conjugales sont trop peu dénoncée est insuffisamment porté à la connaissance de la justice, d'où la nécessité réellement de communiquer à tous les niveaux, d'une certaine manière, tout le monde doit être sensibilisé concernés est aussi responsable d'où la nécessité de privilégier aussi la prévention, c'est souvent rappeler la formation des forces de sécurité, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, je crois que c'est toutes celles qui sont aussi concernés, à ceux la pleine confiance des pouvoirs publics, vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, la politique pénale et puis n'étant Sierre la protéger les victimes, je crois que c'est aussi une des priorités et l'urgence de trouver les bonnes solutions, et je crois que globalement en dont, dans le cas de ma modeste conclusion ce sera surtout faire confiance à la justice par les textes qui vont voir le jour, je crois que c'est aussi une continuité et je crois que c'est, je crois que c'est vraiment une responsabilité de toutes et tous, voilà je vous remercie de votre attention, merci. merci. Voilà, à 17 secondes près, nous sommes exactement dans les temps, mais là, dixit la discussion générale est Close, mais la commission n'ayant pas élaboré de textes, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initial mais Madame Laborde veut prendre la parole, l'auteur de la loi. Merci monsieur le président, vous avez mené ça de main de maître et j'avoue que là, si je peux dire quelques mots, madame Lagarde et sous mes chers collègues, plutôt que cette proposition de loi soit rejetée par l'ensemble des groupes, je préfère demander son retrait, je citerais François Molins, procureur de la République de Paris dans son ouvrage La production judiciaire et médico-légales, pour pénaliser les violences faites aux femmes et protégeant ces derniers en réalité si on ne le fait pas, c'est qu'on n'en a pas la volonté, et peut-être les moyens ajouterais-je ma proposition de loi concerne un trop grand nombre de cas, mais pour bien vous faire comprendre mon incompréhension, quelquefois, je ne comprends pas trop, je vais vous citer un exemple précis, comment peut-on justifier un aménagement des peines quand une personne est condamnée à 3 ans de prison dont 18 mois 18 mois ferme et surtout quand le jugement indiquait en l'état la cour ne dispose d'aucun élément concret permettant d'envisager sérieusement un aménagement de l'emprisonnement, vous comprendrez mon insistance pour toutes ces raisons, malgré tout, et en vous ayant entendu et sachant que mon texte n'est pas mature, du point de vue juridique, je vous demande madame la garde des Sceaux d'être très attentive lors de vos prochains chantiers pour la justice, comme je me permettrai de l'être, en vérifiant si les contenus sont à la hauteur de mes attentes et encore merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette discussion, monsieur le président de la commission des lois, il y aura peut-être une mission sur le sujet que je me permettrai aussi de suivre avec attention, merci à vous tous. Merci. Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 26 du règlement du Sénat l'auteur ou le 1er signataire d'une proposition de loi ou de résolution toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Je peux maintenant un codicille : c'est dans ce cas-là, quelqu'un peut la reprendre, mais la proposition comme il y a plus de temps dans cette niche ça serait inutile, vous êtes complètement informé la séance est levée.

dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit et à 21 heures suite de cette proposition de loi, la séance est levée.